La séance est reprise, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous reprenons la discussion de la proposition de loi relative à l'innovation santé présenté par Madame Catherine Deroche un ni Delmont Koropoulis et plusieurs de leurs collègues, demande de la commission des affaires sociales dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Thomas dessus pour le groupe écologiste pour 5 minutes.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, quel est l'intérêt de ce texte : premièrement, un constat : la France est effectivement en train de perdre sa place dans le développement et la production de thérapies innovantes, les groupes industriels comme Sanofi ou même nos instituts de recherche publique qui, eux, manquent cruellement de moyens non effectivement pas réussi à développer des solutions vaccinales aussi rapidement que d'autres pays, je ne vous refait pas l'histoire, elle est connue et nourrit une petite musique déclinistes qui devient hélas trop familière, la course aux vaccins n'est que la partie émergée de l'iceberg en matière de biotechnologie et de biotech, la France n'est plus à la pointe de l'innovation, c'est vrai, l'un des effets positifs de cette période de pandémie et qu'enfin l'État français prend la recherche médicale au sérieux, il était temps, le gouvernement a investi plus de 7 milliards du plan de relance dans les 2 technologies dans le cadre du plan Innovation Santé 2030, c'est une bonne chose, mais vient alors un autre refrain tout aussi problématique l'innovation médicale deviendrait un enjeu de compétition économique entre puissances scientifiques bien plus qu'un enjeu de santé améliorer le bien-être des individus, que ce soit en France ou à l'échelle mondiale n'est plus qu'un objectif, toujours présent, certes, mais un objectif parmi tant d'autres, je crains que ce soit le modèle qui sous-tend cette proposition de loi ce modèle comporte en lui des évolutions intrinsèque, le patient devient l'agent de sa propre santé et le médecin devient de plus en plus un technicien dans un cadre institutionnel, 2 ans de plus en plus guidés par des impératifs de santé d'efficacité économique et de performance administrative, la logique de soins s'éloigne, ceci étant dit, la médecine personnalisée et les biotechnologies recèle des promesses de progrès médical important pour nos concitoyens ainsi en prenant en compte les caractéristiques bio-génétique génétique et épigénétique dans le traitement de chaque individu, la médecine pourrait réaliser des progrès décisifs dans la lutte contre le diabète, certains cancers ou les maladies génétiques rares, dans ce contexte, comment faire advenir des avances des avancées médicales vertueuse pour toutes et tous, tout d'abord, j'attire votre attention sur le fait qu'acheter des résultats rapides en investissant massivement dans quelques superstars est un leurre, la recherche fonctionne sur le temps long, elle se base sur un travail de fond et sur l'exploration de voix originale qui ne paraissent pas immédiatement porteuse commercialement c'est le b.a-ba de la recherche, elle est aujourd'hui chroniquement sous-financé, dans notre pays, nous ne sortirons pas de l'ornière tant que seuls 2 2 pour 100 de notre PIB sera consacré à la recherche, à titre de comparaison, on est à 3 1 en Allemagne et 2 8 aux États-Unis, la recherche est une affaire de coopération une affaire globale de manière croissante les enjeux de la recherche doivent se penser et doivent être coordonnées au niveau européen pour être réellement efficace, la prochaine étape, et donc, nous semble-t-il, de réussir à coordonner nos plans d'action et d'investissement avec nos voisins européens, je tiens à affirmer dès maintenant l'importance d'une notion clé sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir lors des débats autour des amendements du groupe écologiste, je veux parler de démocratie sanitaire, il s'agit d'une part, de permettre aux citoyens et à la société civile, d'être impliqué dans les prises de décision, d'autre part que les décisions relatives aux soins aux médicaments aux traitements soient prises dans un maximum de transparence, le risque est que la technicisation et la complexification croissante des enjeux liés à la santé fasse perdre confiance aux citoyens dans les mécanismes de décision dans le bien-fondé des décisions prises, nous avons hélas pu le constater ces derniers mois, c'est selon ce prisme que nous abordons ce texte cette proposition de loi essentiellement technique comporte toutefois des avancées indéniables je tiens notamment à saluer le travail de mes collègues concernant les articles encadrant le L7 AFUB voulue par le gouvernement, la sécurisation des données de santé de nos concitoyens, être essentiel en effet réserver l'hébergement et la gestion de ces données à des acteurs européens permet de s'assurer que c'est bien la législation nationale et européenne de protection des données individuelles qui s'appliquent, malgré des différences de fond avec le texte de la commission, force est de constater que cette proposition de loi est un motif d'espoir pour nos concitoyens d'accéder plus rapidement à des traitements innovants, c'est pourquoi le groupe écologiste votera pour l'adoption de ce texte, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à Madame Laurence Cohen pour le groupe CRCE pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé en juin dernier lors de la réunion du Conseil stratégique des industries de santé un plan Innovation Santé 2030, ce sont 7 milliards d'euros qui seront investis d'ici à 5 ans en faveur de la recherche, des industries, des entrepreneurs et des patients sur ces 7 milliards un milliard d'euros sera financé par nos cotisations sociales sur le budget de l'assurance-maladie, ce plan d'investissement intervient après que la pandémie, a mis en lumière les faiblesses de l'industrie pharmaceutique française qui a été incapable de trouver un vaccin contre la Covid 19 ou encore d'éviter les ruptures de stock de médicaments après avoir délocaliser la production en Asie, c'est notamment le cas de l'entreprise Sanofi qui a encore supprimer des postes 364 en recherche et développement en janvier dernier tout en versant des sommes phare unique à ses actionnaires et qui est toujours incapable de produire son vaccin, pourtant c'est son président Olivier Beaud JO que le 1er ministre Jean Castex a chargé de diriger le comité de suivi du plan Innovation Santé 2030, il serait intéressant de savoir quels sont les critères qui sont, qui ont présidé à un tels choix on voit pourtant une nouvelle fois que les logiques de rentabilité de l'industrie pharmaceutique viennent à contre sens de la santé, alors même que les grands labos pharmaceutiques sont redevables en très grande partie des aides financières publiques directes et indirectes la PPL du groupe Les Républicains compile des recommandations formulées par la commission des affaires sociales du Sénat dans ce rapports de juin 2018 sur l'accès précoce aux médicaments innovants et de juin 2021 sur l'innovation en santé elle relaie ainsi les exigences du Lemme Syndicat des entreprises du médicament pour réduire les délais, les contrôles et maximiser les profits au nom du renforcement, je cite, de l'évaluation éthique de la recherche en santé et de l'amélioration des conditions d'accès aux thérapies innovantes, je veux rappeler ici que l'innovation n'existe pas en santé, l'agence européenne du médicament, le dit clairement innovants ne veut rien dire de plus que nouveau cette terminologie est utilisé en réalité en l'absence de nouveautés pour imposer des prix toujours plus élevés face à l'augmentation considérable des prix des nouveaux médicaments, notamment ceux contre le cancer, l'hépatite C et certaines maladies rares, la société civile française se mobilisent pour dénoncer l'opacité des prix, le manque de transparence des négociations entre l'État et les industriels, les répercussions budgétaire et financière, sur l'assurance maladie, ainsi que les conséquences des pénuries de médicaments, elle se mobilise aussi pour améliorer l'accès de toutes et tous aux progrès thérapeutiques, d'autant que des personnes malades, notamment atteints de pathologies orphelines ou en situation d'échec de traitement témoignent chaque jour de besoins thérapeutiques encore insatisfaits et survivent dans l'attente de médicaments efficaces et bien tolérés, si les avancées thérapeutiques sont réelles dans certains domaines, les médicaments apportant une véritable amélioration sont beaucoup moins nombreuses que l'une que les nouveaux médicaments, une étude américaine a ainsi démontré que sur 58 médicaments anticancéreux, entre 1995 et 2013 les médicaments les plus récents n'ont pas augmenté la durée de survie par rapport aux médicaments plus anciens par compte, leur prix a fortement augmenté, plus 12 % par an et dépasser 200000 dollars au nom de l'innovation, les industriels veulent toujours plus, réduire les délais d'évaluation des médicaments au détriment de la lutte contre les conflits d'intérêts et parfois même de la sécurité des patients, il nous semble, à ce propos que la dérogation au système de tirage au sort à l'article 3 peut remettre en cause l'indépendance des comités en créant des risques de conflit d'intérêts par ailleurs les critiques sur les délais d'évaluation des traitements masque mal la partie la plus longue du processus, les négociations tarifaires entre les industriels et le comité économique des produits de santé, notre système de santé permet en réalité déjà des délais rapides de mise sur le marché de médicaments innovants en ayant recours par exemple aux autorisations temporaires d'utilisation qui existe depuis 1994 cette PPL propose également de modifier les critères de fixation des prix, en ayant recours aux critères de la valeur de la valeur thérapeutique relative ce mécanisme existe déjà sous l'appellation contrats de performance dont la Cour des comptes dressait un bilan accablant, en 2017 plutôt que de permettre aux Start-Up, aux laboratoires de renforcer leurs marges financières, comme le propose cette PPL il est urgent de retrouver une maîtrise publique dans la politique du médicament et de socialiser tout en partie ou partie des firmes de la Big Pharma afin de créer un pôle public industriel en France et en Europe, c'est le sens de la proposition de loi portant création d'un pôle public du médicament et des produits médicaux déposés par notre groupe et, malheureusement, rejetée par le Sénat en décembre 2020 et que nous n'avons pas pu présenter en amendement du fait de l'Arctique 40 pour l'ensemble de ces raisons, les parlementaires du groupe communiste républicain citoyen écologistes voteront contre cette proposition de loi, je vous remercie. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission madame la rapporteure, mes chers collègues, je ne suis ni médecin ni chercheur ni biochimiste, aussi ai-je fait un atterrissage un peu brutal en abordant la PPL proposée par Catherine Deroche et Annie Delmont Koropoulis au fil des lectures et des auditions, je me suis trouvé d'abord perdu au milieu d'acronymes nouveau moi qui maîtrise, surtout ceux de l'affaire des collectivités territoriales, cette phrase de Barjavel mais même revenu en mémoire tant qu'on a essayé de combattre la peste avec des mots latins, elle a tranquillement dévorer l'humanité, mais j'ai vite saisi l'essentiel pour retrouver son rang mondial dans le développement et la production de thérapies innovantes, la France a besoin de fluidifier et simplifier et rendent plus opérationnels tout l'écosystème de la recherche en santé désormais ces préoccupations ne sont plus le seul apanage des experts car la pandémie a mis les sciences biologiques et de santé au centre des préoccupations de tous les Français la crise sanitaire a été à la fois un accélérateur puissant d'innovation, mais aussi un révélateur de l'état inquiétant de la dispersion des moyens et de la complexité de l'organisation du fonctionnement et du financement de la recherche en général, mais plus particulièrement de celle en biologie santé et je cite ici un rapport de l'Académie de médecine, l'article 1er vise à autoriser à autoriser le déploiement d'essais cliniques au domicile des patients, il suffit de penser aux difficultés logistiques pour les malades atteints de pathologies rares, en particulier les enfants pour se rendre vers les centres spécialisés pour mesurer l'intérêt majeur d'une telle avancée : l'évaluation de l'éthique des recherches sans alourdir pour autant les procédures est au coeur de cette PPL les CPP deviendront donc, selon l'article 2 des comités d'éthique de la recherche et de la protection des personnes, il est proposé une refonte importante des comités de protection des personnes, leur nom, leur composition, leur rattachement systématique à un CHU ou tout autre établissement de santé d'intérêt collectif afin de rétablir la continuité de la recherche fondamentale jusqu'à la recherche clinique, la création d'un référentiel d'évaluation, l'établissement d'un cadre convergents qui permettent à la fois de les rendent plus opérationnels et de valoriser les missions des universitaires et praticiens hospitaliers qui s'y investissent, selon les données de la direction générale de la santé, le délai médian global d'autorisation des essais cliniques de médicaments, tous domaines confondus, s'établit à 77 jours sur les 3 premiers mois de l'année, de 2021 les CPP, au nombre de 39 sur le territoire ne dispose pas des moyens humains, financiers et techniques permettant d'absorber leur charge de travail, ils sont eux en Bolivie cette PPL ouvrent des pistes pour y remédier, il me semble que c'est essentiel car en reprenant ma vision de béotien que je ferai à ce sujet, 3 constats : le 1er c'est que pour certains patients 77 jours ça peut être vitale et je pense ici à Camille, qui a tant espérer accéder à la thérapie expérimentale de la dernière chance, le second c'est que nous traversons une crise sanitaire majeure qui nous a fait collectivement mesurer toute l'importance de chaque jour qui passe, le 3ème, c'est que les groupes pharmaceutiques privilégieront pour leurs essais cliniques, les pays où les délais seront les meilleurs le chapitre 2, tend à favoriser le développement de la recherche dans le domaine de la médecine dite personnalisée, celle des 5 p préventive prédictive personnalisée participative et de preuves, je laisserai ma collègue Jocelyne Guidez et des titres de et vous aurez compris mes chers collègues, que l'Union centriste soutient soutient ces dispositions qui doit permettre d'améliorer tant la souveraineté et la sécurité sanitaire que la qualité de vie des patients plus que tout, nous aider à sortir d'un carcan administratif qui ne cesse de croître, faire sauter les tuyauteries et peut-être conclure comme Camus et un avec un peu d'amertume, la seule façon de mettre les gens ensemble, c'est encore de leur envoyer la peste. peste. Bon, vous oubliez Madame Sollogoub quand je préside éviter de nous envoyer des maladies parce qu'elle est la parole est maintenant un Madame Véronique Guillotin, pour le groupe RDSE pour 5 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, madame la présidente de la commission, chers collègues, la proposition de loi que nous allons examiner, a le mérite de s'attaquer à des sujets qui s'apparentent à des sujets d'initiés, mais qui ont pourtant des conséquences sur la vie et la santé de bon nombre de Français en pointe sur ce sujet, grâce à de son dispositif d'autorisation temporaire d'utilisation la TU La France a permis dès les années 90 un large accès accès de patients atteints de maladies graves à de nouveaux médicaments avant leur autorisation de mise sur le marché des avancées sont également à saluer lors du CSIS, 2021, mais le chemin à parcourir reste encore à faire, afin, j'y arriverai, excusez-moi, afin que l'ensemble des besoins thérapeutiques urgent accompagné avec souplesse, l'innovation à maintenir l'attractivité de la France sur une scène internationale de plus en plus concurrentiel concurrentiel et je pense que il est important de le redire également cette proposition de loi fondée sur 2 rapports auxquels j'ai collaboré avec mes collègues Annie Delmont Koropoulis et Catherine Deroche cherche à y apporter des réponses, je salue l'excellent travail qui a été réalisé par la rapporteure, c'est un travail difficile technique de qualité menée à l'issue de nombreuses auditions. Aussi, nous soutenons l'esprit général de ce texte que l'examen en commission a permis d'enrichir l'article 1er va faciliter le déploiement d'essais cliniques en ambulatoire en autorisant, qu'ils soient réalisés au domicile des patients rendant également possible la télémédecine les CPP qui vise à s'assurer que toutes les recherches impliquant la personne humaine en France respectent des exigences médicales éthiques et juridiques seront renommés, comité d'éthique de la recherche et de protection des personnes, c'est RPP pour mieux coller à la fois leur mission et à ce qui se fait dans la majorité des pays européens à travers les articles 3, dit ce texte entend octroyer au RPP, plus de moyens, précise les modalités de contrôle par les ARS et propose des mesures renforçant l'attractivité des fonctions de membre du CE RPP, en accord avec l'amendement que j'avais déposé en commission le rattachement DCRTP à tout établissement de santé d'intérêt collectif répond à une demande forte des établissements, y compris des instituts pour le cancer, donc tout cela va dans le bon sens, l'article 6 un peu plus épineux tente de répondre à l'engorgement des CPP par les projets de recherche impliquant la personne humaine R il y a chaîne 3 la solution retenue par la rapporteure de faire appel si besoin au comité d'éthique de la recherche par une solution souple et adaptée, j'ai bien compris que des désaccords existaient sur ce point, la 2ème partie de la proposition de loi vise à améliorer l'accès des patients aux innovations, la mesure phare est la création d'un forfait de caractérisation d'un cancer, permettant ainsi de prendre en charge la recherche de biomarqueurs diagnostiques pronostic ou Hanno Stick pour tout nouveau cancer diagnostiqué chez un patient je présenterai 3 amendements cet article 14 j'ai en effet été alerté sur les risques potentiels d'une telle mesure, si elle était adoptée en l'état, la prise en charge est très variable d'un cancer à l'autre, d'une région à l'autre, il est également habituel que le diagnostic soit effectuée par étapes dans plusieurs établissements, sur demande de prescripteurs différents, y compris après un geste chirurgical ou l'échec d'une première ligne thérapeutique pour être pleinement efficient, ce forfait doit donc être suffisamment souple pour être utilisés à différents moments du parcours du patient à partir du diagnostic, le cas particulier de la récidive mérite également d'être précisé les articles 16 à 18 Vienne simplifier la prix du fixation du médicament, accélérant ainsi l'accès des patients aux médicament innovant dans le cas où l'amélioration du service médical rendu est difficile à mesurer, c'est le critère de valeur thérapeutique relative qu'il en faudra le prix les donner envie réelle seront mieux prises en compte et on revient effectivement à l'aspect concurrentiel qu'il existe au niveau de nos pays, enfin, je profite de cette tribune, Madame la Ministre, pour évoquer la nécessaire réforme du référentiel des actes innovants hors nomenclature l'oreille créée en 2015 pour permettre une prise en charge temporaire et dérogatoire des actes innovants depuis 2018 les tests génétiques sont remboursés à l'établissement prescripteurs via une enveloppe nationale malheureusement fermé, or le volume des tests effectués en constante augmentation, ce qui devrait être une bonne nouvelle puisque les patients accèdent ainsi à une prise en charge personnalisée se transforme en fait en casse-tête financier pour les établissements qui supporte 100 % des coûts mais n'en sont remboursés qu'à hauteur de 47 le reste à charge pour un établissement peut atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros par an, puisqu'il est question de l'excellence de la médecine française de sa souveraineté et de l'amélioration de l'accès des patients aux innovations, nous pensons que ce frein doit être rapidement levé, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à Madame Émilienne Pommerol pour le groupe socialiste, pour 9 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, nous sommes appelés aujourd'hui à nous exprimer sur la proposition de loi de Madame, la présidente de la commission des affaires sociales, donc madame de roches et de Madame Delmont Koropoulis se portant sur l'innovation en santé au vu de son titre du nombre de ces articles, encore plus après lecture des 2 rapports parlementaires très fouillée relatives aux médicaments innovants de licencier s'inspirer, c'est un petit peu un sentiment d'inachevé qui prédomine à l'époque de la santé globale et de la médecine des quatre P. quand on parle d'innovation, de santé, on s'attend à ce qu'il soit question certes de médecine personnalisée qui est abordé ici, mais sous un angle purement déclaratif mais également de médecine préventive prédictive et participative, ainsi bien sûr que l'enjeu de la santé environnementale, mais le texte présenté aujourd'hui presque exclusivement fondre focalisé sur l'innovation thérapeutique, voire médicamenteuse à partir de ce phase clinique, qu'un article par exemple sur la recherche fondamentale, pourtant à l'origine de l'innovation, très souvent, comme nous l'avons vu lors de la crise du du Covid 19 le développement des vaccins à ARN repose sur des années de recherches précédentes dans ce domaine, impossible non plus de ne pas relever que l'accès aux médicaments innovants ne cesse de faire l'objet de modifications législatives depuis plusieurs le PLFSS avec l'entrée en vigueur en juillet dernier de l'accès précoce qui avait été voté dans le lot de finances 2021 et l'adoption sur la loi de finances devait de 2022 en décembre dernier, le dispositif expérimental d'accès Direct, donc non encore mises en oeuvre ici la majorité sénatoriale psy prompte à définir à défendre à la prévisibilité pour les entreprises, notamment en matière fiscale, ajoute sa propre Pierre à système dit-il législative qui est problématique quand elle l'adaptation des acteurs de la filière industrielle du médicament et à l'absence de visibilité indique pour eux et ce d'autant plus que dans le domaine des biotechs, on a surtout à faire à des Start-Up et des PME, pour lesquels la visibilité est encore plus importante, 3 volets dans ce texte, donc 2 pourrait avoir une portée très pratique, celui sur les comités de protection des personnes CPP et celui sur l'expérimentation de nouveaux critères de fixation des prix des médicaments innovants concernant le 1er volet le texte s'attache à rénover les conditions de validation éthique des projets de recherche impliquant la personne humaine à travers le fonctionnement des CPP, qui est une question récurrente depuis plusieurs années leur dimension éthique et réaffirmé ce qui était minimum positif à accorder à cette proposition de loi, de même que le portail unique de soumission des projets de recherche, elle répond également à la demande des associations de patients, de constitution d'une liste d'experts pour répondre à l'enjeu des compétences de plus en plus pointue qu'exige l'évaluation des projets de recherche en revanche le rattachement CPP CHU et de nature à remettre en question leur indépendance, c'est un point de divergence, pour nous, l'indépendance des CPP constituant le fil rouge notre positionnement sur ce vol, texte nous avons d'ailleurs déposé un amendement dans ce sens, nous estimons que les dysfonctionnements de l'évaluation éthique de la recherche biomédicale pose avant tout la question des moyens à la disposition des CVP pour remplir leur mission et au caractère bénévole de leurs nombres qui impacte leur disponibilité, la loi de finances de 2021 à augmenter la contribution sur le chiffre d'affaires des industriels pharmaceutiques afin d'attribuer le rendement c'est supplémentaires ainsi obtenues au CPP, quelle est l'émission de cette mesure est-elle suffisante pour l'instant nous n'en savons rien et c'est dommage, concernant le second volet, la proposition de loi ont ont accéder à une demande récurrente de l'industrie du médicament, la prise en compte de la valeur thérapeutique relatif dans la fixation du prix des médicaments dits innovants et présentant, je cite, une efficacité, une sécurité pouvant être présumé et répondant à un besoin thérapeutique majeur au au regard des alternatives existantes, vous connaissez notre attachement au groupe socialiste, écologiste et républicain au principe de transparence du prix des médicaments et du prix juste équilibré entre le triptyque bénéfice pour la santé publique, coût pour la société et la protection sociale et enjeux industriels, or le dispositif telle qu'il nous est proposé ne répond pas à ces considérations, nous aurons donc des propositions en ce sens à l'article 16 dans ces derniers articles, textes abordent le sujet de la plateforme lui donner en de santé World qui est un enjeu majeur pour l'avenir de notre système de santé car c'est bien la question de la gouvernance éthique des données massives de santé de nos concitoyens qui est posée, et force est de pointer le manque de garanties qui risquent d'obérer sérieusement non seulement sa mise en Oeuvres mais également l'acceptabilité sociale de celle-ci, face au risque de fuite de ses données très sensibles d'ailleurs le gouvernement lui-même a été obligé de mettre un coup d'arrêt à son déploiement avec le retrait de sa demande d'autorisation auprès de la CNIL, la centralisation du système national des données de santé dans la plateforme des données de santé dans ces conditions nous souscrivons totalement à l'objectif de sécurisation du stockage des données de santé en réservant leur hébergement et leur gestion à des opérateurs relevant exclusivement de la juridiction européenne je terminerai mon propos n'évoquant de certains sujets qui nous sommes, devoir être pris en considération dans le domaine de l'innovation suite à quelques conditions auxquelles j'ai participé de travaux menés par ailleurs par la mission d'information sur la sécurité sociale, environnementale du XXIe siècle qui a été initié par le groupe écologiste sociale l'hilarité et territoires, nous sommes que nous devons partager le constat dressé par la rapporteure, qu'il y a une nécessité à réformer transformer notre système de santé notamment en prenant en compte la question de la prévention. Construit après la Seconde Guerre mondiale, notre système et nos politiques de santé sont ne sommes très sur le traitement des patients et exclu son environnement social et les déterminants sociaux de son état de santé, l'environnement familial, le vide, ville, niveau d'éducation etc en se centrant sur le patient et la maladie, le système de soins s'est détourné de la définition de la santé, porté par l'OMS, non plus comme une absence de maladie, mais comme un état complet de bien-être physique, mental et social, il apparaît donc indispensable de concevoir des politiques de santé fondée sur la valorisation de la bonne santé, cela implique de sortir du modèle uniquement curatif et de s'intéresser à la question de la prévention et l'éducation à la santé, le texte évoque sans le développer, nous le regrettons la notion d'Expo somme il est désormais établi que notre santé dépend une grande partie de l'homme drôlement dans lequel nous évoluons les facteurs environnementaux seraient à l'origine de plus de 70 % les maladies chroniques non transmissibles qu'il s'agisse de pathologies cardiovasculaires métaboliques, cancers ou autres respiratoires, problèmes respiratoires chroniques, il apparaît aujourd'hui qu'il serait indispensable d'étudier non plus l'effet sur la santé humaine de chaque facteur incriminé séparément mais plutôt dans leur ensemble, il y en effet quand certains agissent en synergie, d'autres peuvent se compenser avec une bonne connaissance des exposants et de leurs impacts on pourrait non seulement prédire. Des risques de santé, de manière à proposer des prise en charge précoce aux personnes concernées mais aussi agir pour tendre vers que nous sommes les plus favorables possibles à notre santé et à notre bien-être, cette question pose également celle de la transversalité du décloisonnement dans nos réflexions sur la santé humaine, la santé environnementale et la santé animale. Développé, donc par le concept One s, il apparaît désormais primordial de s'interroger sur la place de la santé, l'homme d'autres politiques publiques c'est réel, l'alimentation, la santé au travail, la santé scolaire le modèle énergétique, la pollution de l'air et de mettre en place une meilleure coordination entre les ministères, notamment ceux de la santé de la transition écologique ou de l'agriculture, vous l'aurez compris mes chers collègues, si nous partageons l'objectif bien sûr d'améliorer l'innovation en santé, notre position globale notre positionnement global sur cette proposition de loi sera déterminé par le sort réservé dans la discussion à nos amendements, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à monsieur Martin lévrier pour le groupe RDPI pour 6 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, mes chers collègues, des premières découvertes de l'institut Pasteur au coeur Carmat Le coeur artificiel le plus avancé au monde produit dans les Yvelines, la France ouvre régulièrement la voix pour mieux soigner depuis près d'un siècle et demi je souhaite d'ailleurs prendre ce temps pour saluer la mémoire de François Gros, co-découvreur de l'ARN messager précurseur, précurseur du séquençage et de la cartographie génétique décédé la semaine dernière, nous devons à ces chercheurs à ces passionnés du progrès au service de l'humain, de lever les barrières existantes pour permettre des découvertes essentielles pour autant, force est de constater que la crise sanitaire a constitué un épisode douloureux pendant lequel notre pays a dû prendre la mesure de certaines de ses faiblesses dans le domaine de la santé, c'est pour rappeler l'impérieuse nécessité de donner un nouvel élan à l'innovation et de travailler en synergie sur ces sujets que vous avez lancée en juin dernier Madame la présidente de la commission des affaires sociales, une mission flash près Conseil stratégique des industries de santé dans le but de dresser le bilan de la mise en oeuvre des mesures du 8ème CSIS et préparer le suivant le préparer

c'est dans la même logique, madame la présidente, que vous avez déposé le 25 novembre 2021 aux côtés de Madame la rapporteure Annie Delmont Koropoulis et plusieurs de vos collègues cette PPL dans le but de renforcer l'évaluation éthique de la recherche en santé d'améliorer les conditions d'accès aux thérapies innovantes et de renforcer l'usage sécurisé des données de santé, ce texte comporte 23 articles qui s'inscrivent dans le contexte d'un soutien à l'innovation et à la sécurité d'approvisionnement engagée par le président de la République, avec notamment le plan Innovation Santé 2030, qui assurera l'émergence de véritables champions français dans le domaine de la santé, ce plan Innovation Santé 2000 tranches engage 7 milliards d'euros, un milliard pour le renforcement de la capacité de recherche biomédicale 800 millions dans la biothérapie et la bioproduction de thérapies innovantes 650 millions pour la santé numérique 3,5 milliards pour le soutien à l'industrialisation des produits de santé sur le territoire français, sans oublier la création d'une structure d'impulsion et de pilotage stratégique, stratégique de l'innovation en santé avec l'agence d'innovation de santé. Renforcer la souveraineté française en prenant les virages des biotechnologies et on accompagnant davantage les biotechs françaises, faire de la recherche, un objectif majeur de santé publique : lever les freins dans l'accès précoce aux médicaments et aux traitements innovants, passer de la médecine curative à la médecine prédictive en valorisant les données de santé sans négliger l'encadrement de leur utilisation, anticiper les maladies infectieuses émergentes, voilà les étapes indispensables qu'il nous faut franchir si nous voulons permettre à la France de rester pionnière en santé publique votre texte, madame la présidente, propose ainsi des améliorations bienvenues tels que, à l'article 1er la possibilité de réaliser des recherches au domicile de participants ou encore l'insertion du mot éthique dans les comités de protection des personnes, nous nous félicitons également de l'introduction, l'article 10 bis qui reprend une mesure de nôtre que l'autre groupe avait tenté d'insérer dans la loi bioéthique, afin de simplifier les démarches des promoteurs ayant obtenu une autorisation de l'ANSM ou d'un CPP grâce au travail remarquable de Madame la rapporteure certaines limites que nous avions constaté dans la rédaction initiale ont déjà été résolus lors de l'examen en commission, je pense notamment à la suppression de la vie de de l'ANSM dans le cadre de l'agrément d'un CPP par le ministre chargé de la santé, pour autant, certaines limites demeurent et nous invite à une certaine réserve, c'est le cas d'missions de prospective, de veille et d'évaluation donnée à l'achat à la HAS pour les dispositifs les plus innovants sur le fond, nous accordons sur l'importance d'un telle rôle pour rester au 1er plan de la recherche dans le domaine de l'état de l'innovation en santé mais cette mission sera au coeur de la mise en place de l'Agence de l'innovation en santé et il semble préférable de ne pas légiférer avant l'institution de celle-ci, il en va de même pour les articles sur les données de santé, là encore, nous partageons l'objectif affiché, les données sont une source de valeur ajoutée unique qu'il ne faut mais mais il n'apparaît pas nécessaire aujourd'hui de légiférer sur des mesures qui sont satisfaites à l'instar du traitement de données des organismes complémentaires, ou sur le point de l'être, je pense ainsi à l'hébergement de données au niveau européen, enfin, de nombreuses mesures sont proposées en parallèle d'un large mouvement engagé au niveau national par le gouvernement à travers le plan Innovation Santé 2030 et au niveau européen, je pense par exemple au règlement sur l'évaluation des Technologies de la santé, adoptée par le Parlement européen en décembre dernier après plus de 3 ans de travail la temporalité questionne et crée un risque de redondance, vous l'aurez compris, bien que nous accordions sur l'objectif affiché pour la pour assurer à la France un rôle à part entière dans cet écosystème nous demeurons plus réservé sur certains des moyens présentés pour y parvenir, et je le redis, sur la temporalité du texte, c'est pourquoi notre groupe s'abstiendra mais nous luttons pas que la navette parlementaire sera l'occasion d'enrichir ce texte, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à Madame Vanina Paoli pour le groupe, les indépendants pour 5 minutes.

madame la ministre, mes chers collègues, le 22 février 1942 il y a 91 ans jour pour jour, Stéphane Schleck mettait fin à ses jours à Petropolis, au Brésil, l'auteur du Monde d'hier, qui a grandi dans le rêve d'une Europe pacifique ne supportait plus le spectacle atroce d'un monde en guerre, quelques années plus tard, après toutes ces horreurs, le grand projet européen prenait vie pas, il aurait sans doute adhérer à cette grande entreprise de paix, de tolérance et de prospérité. 80 ans plus tard, après 2 ans de crise sanitaire, nous savons que le virus a profondément bouleversé le cours de l'histoire, mais nous ignorons encore précisément en quoi le monde hier tranchera avec le monde de demain dans ce contexte, encore très confus, nous pouvons toutefois d'ores et déjà identifié quelques priorités politiques au moins 2 me paraissent essentiels : la première, c'est l'urgence pour l'Europe et plus encore pour la France de recouvrer sa souveraineté sanitaire on se réindustrialiser, nous avons pris conscience au début de l'épidémie de la situation de dépendance dans laquelle notre pays se trouver cette situation n'était pas nouvelle, loin de là, elle s'était installée progressivement à mesure que trop d'élite, trop de grands patrons ont fait leur la théorie mortifère de la France, sans usine, conforté par des gouvernements qui ont prioriser le tout cols blancs et le bac pour tous, peu à peu les usines fermées, nombre de nos ingénieurs et de nos chercheurs, quitter le pays, cette croyance notre supériorité ce refus de regarder la situation avec lucidité laisse pantois : la prise de conscience au printemps 2020 n'en fut que plus brutale, peu à peu, nous avions abandonné des pans entiers de notre appareil productif, nous réalisions qui avec ce démantèlement, nous ne pouvions plus produire ni masque, ni médicaments, surtout au pays de Pasteur notre incapacité à développer un vaccin contre la Covid nous a fait acter une forme de déclassement scientifique et industriel, la seconde priorité découle directement de la première, c'est la nécessité pour la France de revenir à la pointe de l'innovation santé en la matière, il s'agit, à mon sens, moins de miser sur la recherche fondamentale que de renforcer notre capacité à convertir convertir nos savoirs fondamentaux en solutions industrielles, la tâche est immense, nous devons nous y atteler au plus vite pour espérer des résultats à moyen terme, c'est pourquoi je me réjouis que le Sénat s'empare de ce sujet, bien sûr, il n'est pas possible dans traités par dans tous les aspects dans le cas d'une seule proposition de loi dont je salue les auteurs mais face à l'ampleur de la question, je doute que la réorganisation des comités de protection des personnes qui occupera une part importante des discussions constituent une vraie priorité d'action pour faire de la France, la terre de l'innovation santé à mon sens, il est beaucoup plus urgent de créer les conditions d'émergence et de consolidation d'écosystèmes d'innovation performant pour ce faire, la collaboration entre acteurs publics et privés est essentielle, elle doit soutenir une approche de la recherche, fondée sur une confiance partagée, cela implique notamment de faire évoluer les modèles financiers afin de permettre aux entrepreneurs de développer de nouvelles solutions sans être contraint par des délais raccourcis, de retour sur investissement, il s'agit de renouer avec le temps long, de la recherche qui est l'une des conditions indispensables pour générer l'innovation de rupture et le changement structurel mais tant l'on ne signifie pas allongement des procédures forte au contraire puisque les innovateurs doivent pouvoir se consacrer pleinement à leur recherche sans pression d'une rentabilité à court terme ni procédures administratives chronophages, notre devoir, mes chers collègues et de leur faciliter la tâche, l'objectif est donc en toute sécurité évidemment de simplifier au maximum l'accès au marché, c'est pourquoi je me réjouis que le texte consacre plusieurs articles à l'amélioration et à l'ouverture du système national des données de santé : la possibilité pour les entreprises innovantes, d'utiliser les données vie réelle doit permettre de faire évoluer en profondeur les modèles économiques, concrètement, cela permettra de basculer une partie des délais incompressibles de la R&D sur l'aval de la mise sur le marché plutôt que de tout concentrer sur l'amont, l'idée est de mieux articuler 2 impératifs de l'innovation, à savoir d'une part la nécessité du temps long, et d'autre part la nécessité la nécessité, pardon, de l'itération et de l'amélioration constante, par ailleurs, cette évolution ouvrent d'autres champs d'investigation, tels que la protection des données et de suivis en vie réelle des effets des médicaments, nous n'aurons pas le temps de traiter tous ces sur tous ces sujets, mais le texte que nous allons examiner nous permet déjà de proposer quelques pistes d'action concrète et pour ma part je vous proposerai quelques moment ce sens notre groupe les indépendants républiques et territoires votera en faveur de ce texte, je vous remercie. Merci, cher collègue, la paix, la parole est maintenant à Madame Florence Lasserre a, pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis ce soir pour examiner la proposition de loi relative à l'innovation santé présenté par nos collègues Catherine Deroche et Annie Delmont groupe glisse cette proposition de loi s'inscrit dans le prolongement des recommandations formulées par la commission des affaires sociales dans ses rapports sur l'accès précoce aux médicaments innovants et sur l'innovation en santé, elle a pour objectif de renforcer l'évaluation éthique de la recherche en santé et d'améliorer les conditions d'accès aux thérapies innovantes, la crise sanitaire, a rappelé l'importance du secteur de la santé comme un élément stratégique de souveraineté sans conteste l'absence de vaccin au pays de Pasteur et le symptôme de ce qui s'apparente à un déclassement de notre pays dans le développement et la production de thérapies innovantes, force est de constater le constant recul de la France dans le domaine de la recherche médicale et d'innovation, passant en terme de production de publication de la 5ème place en 2000 à la 6ème en 2010 et à la dixième depuis 2019, comment expliquer cet effacement progressif depuis 2011 les crédits publics pour la recherche ont baissé de 28 % mais l'aspect budgétaire n'explique pas tout, une action uniquement budgétaire ne suffira pas à elle seule pour permettre à la France de disposer d'une recherche forte dans le domaine de la santé, il existe en France une forte dynamique des entreprises du secteur de la santé, en revanche, il manque une coordination entre cette dynamique et la capacité de notre système de soins et de l'ensemble des acteurs des autorités sanitaires à accompagner l'innovation santé d'autre part, innovation ne peut se concevoir qu'en remplaçant le patient au coeur du dispositif, les patients doivent avoir accès rapidement aux innovations, ce texte propose quelques solutions, il est tout d'abord nécessaire de réunir les conditions d'un développement de la recherche en santé, c'est l'objectif du tri trop 1er de cette proposition de loi qui ambitionne de rénover l'évaluation éthique de la recherche en santé, l'article 1er vise ainsi à faciliter le déploiement d'essais cliniques en ambulatoire en autorisant la réalisation au domicile des participants aux recherches et en permettant aux promoteurs de désigner des investigateurs chargé de coordonner la recherche par-ci, territoire plutôt que par lieu, l'article 2 renomme les comités de protection des personnes afin d'introduire la notion d'éthique dans leur dénomination conforte conformément à ce qui se pratique chez nos voisins, l'article 3 propose de rattacher systématiquement les comités de protection des personnes, un centre hospitalier universitaire afin de garantir au CPP, les moyens matériels nécessaires à l'exercice de leur mission : cet article prévoit également la spécialisation de certains CPP en pédiatrie et maladies rares, il s'agit de compétences spécifiques dans la bonne identification permettra de soutenir le développement des recherches, les articles 11 à 13 vise à faire du développement de la médecine personnalisée un objectif commun aux politiques de recherche et de santé publique, l'article 14 introduit un mécanisme original visant à mieux prendre en charge le diagnostic d'un cancer, la dernière partie du texte est relative aux données de santé, les données sont un enjeu majeur d'évaluation des médicaments et des dispositifs médicaux car elle permettent un suivi en vie réelle en 2019 le ES Data Hub a été créé, il est chargé de regrouper toutes les données de santé française, l'article 20 de la PPL prévoit d'intégrer dans les finalités du l'évaluation de l'efficacité envie réelle de traitement. L'analyse de ces données contribuera à évaluer les innovations leur intérêt pour les patients, pour que l'exploitation des données soit efficace, il faut que les chercheurs puissent disposer des données à jour afin de mieux rendre compte : l'État français, l'état de santé des Français et de leurs besoins médicaux. Concernant le sujet sensible et données de santé, il est également essentiel de sécuriser l'exploitation des données, 6 mois après la création du Health Data, l'hébergement des données a été confiée par le gouvernement est sans appel d'offres à la plateforme Microsoft multinationales américaines, soumises aux lois extraterritoriales américaines notamment au cloud Act, qui oblige les entreprises américaines ou opérant aux États-Unis à communiquer les données à l'administration américaine, même si celles-ci ne sont pas stockés sur le sol américain ou ne concerne pas le citoyen américain, je me réjouis donc les articles 21 et 22 renforce les garanties des patients, quant à l'usage de leurs données personnelles de santé ainsi l'article 21 interdit l'usage de ces données par les organismes complémentaires à des femmes de sélection des risques et l'article 22 vise sécurité le stockage de données en santé, en réservant leur hébergement et leur gestion à des opérateurs relevant exclusivement de la juridiction de l'Union européenne, ce texte porte des avancées majeures pour l'innovation en matière de santé l'accès des patients aux traitements innovants et la protection des données, de France, je vous remercie de votre attention. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à Madame Jocelyne Guidez pour le groupe Union centriste pour quatre minutes.

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, la présente proposition de loi relative à l'innovation santé a été déposée au Sénat par la présidente Catherine Deroche la s'inscrit dans le prolongement des recommandations formulées par la commission des affaires sociales depuis 2018 je suis particulièrement le rapport d'information sur la refondation de l'écosystème français et européen de l'innovation en santé présenté en juin dernier par nos collègues Annie Delmont Koropoulis et Véronique Guillotin, je tiens à les remercier pour leur engagement dans l'organisation de nombreuses auditions cette porté sur un texte au contenu dense qui, pour des non-espère que moi et très technique, la compréhension des abréviations PS NDS ANSM sécheresse AMM H. et caetera exige une formation de vulgarisation scientifique, néanmoins, nous savons tous que ce texte s'inscrit paradoxalement dans une démarche de simplification des procédures d'accès des patients aux médicament aux force est de constater que le retard français significative dans le développement et la production des thérapies innovantes, malgré les efforts déployés en matière académique industriels et de recherche afin de reconstruire notre appareil d'innovation en santé, cette proposition de loi mérite d'être prises en considération, puisqu'elle entend renforcer l'évaluation éthique de la recherche en santé, améliorer les conditions d'accès aux thérapies innovantes et faciliter le déploiement de ce cliniques, nous ne pouvons qu'apprécier la contribution de la politique nationale de recherche à l'amélioration de la qualité de vie des patients et au renforcement de la souveraineté et de la sécurité ça ne sanitaire, l'adaptation des actions de prévention et des stratégies diagnostique et thérapeutique aux spécificités des patients constitue également une avancée importante, nous saluons l'introduction dans ce, dans le code de la santé publique et du concept de médecine personnalisée, ce texte prévoit en effet d'intégration dans la stratégie nationale de recherche d'un volet relatif à la recherche une novation thérapeutiques incluant un programme dédié à la médecine personnalisée en coordination avec la politique de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation en ce qui concerne l'accès aux patients aux médicament innovant dans l'attente de données cliniques suffisante et pertinentes pour l'évaluation de l'amélioration du service médical rendu par les médicament présentant une efficacité et répondant à un besoin thérapeutique majeur au regard des alternatives existantes, voici ce qu'il y ait accès. ce qui est proposé la fixation du prix de ce médicament pourra tenir compte à titre expérimental, pour une durée de 5 ans d'une évaluation par la Haute autorité de santé de sa valeur thérapeutique relative, en outre, l'évaluation de l'amélioration du service médical rendu des médicaments innovants tient compte des données envie réelle en complément des résultats des essais cliniques, des industriels, s'agissant des données de santé les titulaire d'une autorisation de mise sur le marché ou les exploitants d'un traitement pour évaluer son efficacité en vie réelle peuvent accéder sans sous certaines conditions aux données de santé du système national des données de santé afin de mieux encadrer cet accès, l'article 20 le conditionne à la remise annuelle à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d'une étude dévalant les effets de la prescription des produits, à savoir la tolérance du patient et l'efficacité de traitements, ce dispositif a été complété par un amendement de notre collègue rapporteur conditionnant l'accès de à ces données sensibles mais précieuse à la validation d'un protocole de recherche par le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé cet encadrement nous sommes nécessaires, enfin le texte renforce de garanties des citoyens patients quant à l'usage de leurs données personnelles de santé et interdit l'usage de ces données par les organismes gérant les complémentaires à des fins de sélection des risques, l'article 22 sécurise aussi le stockage de données en santé, en réservant leurs hébergements et leur gestion à des opérateurs relevant exclusivement de la juridiction de l'Union européenne innovation santé devrait être aussi encourager pour toutes les pathologies compris la maladie de la haine et les maladies rares du système immunitaire, enfin, cette proposition de loi vise à résoudre des problèmes existants, il s'agit d'un ajustement qui va dans le bon sens, comme l'a dit ma collègue, Nadia Sollogoub, l'Union centriste votera ce texte, je vous remercie de votre attention. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à monsieur Bruno Belin pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, madame la présidente, madame la rapporteure, mes chers collègues. Plus que jamais, la crise a révélé que se soigner et le 1er, sujet de préoccupation, le 1er, sujet d'actualité, et peut-être le 1er sujet de discrimination, elle a aussi permis de révéler un certain nombre de nouvelles méthodes, parce que la crise a tout chamboulé. Tout à l'heure votre collègue, secrétaire d'État, Take a expliqué que la téléconsultation avait été une solution innovante. Mais il y a pas plus injuste parce que la différence sur les territoires est complètement inacceptable, vous avez des lieux où la téléconsultation est possible Madame la Ministre, faut-il encore que la fibre arrive et puis il y a des lieux où il manque les équipements et donc il faudrait un plan déjà rien que sur ce sujet-là pour accélérer la fibre accélérer la formation soutenir financièrement les installations car si on veut que ça soit une solution, il faut qu'elle soit de même accès pour tous les habitants de ce pays, la crise a révélé 2 choses et je profite de cette tribune pour le rappeler parce qu'elle me semble essentielle certains manquements et je ne parle pas du curare ou des masques de personnes imaginait avoir à utilisé en excès, comme on le fait depuis des mois, je parle de produits tout à fait baptiser que je veux parler du zone ou de certains celle d'aspirine qui ce matin encore manqué en officine alors qu'ils ne coûtent que quelques dizaines d'euros. Et puis elle a révélé surtout un manquement en termes de moyens humains, nous en avons tous conscience parce qu'on a tous le retour dans nos quartiers, ou sur nos territoires ruraux, manque de moyens et donc. Avant de se préoccuper des solutions Data 3,0. Au tout numérique, rappelons-nous que rien dans le diagnostic ne remplacera l'écoute, l'humain, avec ce regard de l'environnement qui peut évidemment concerné demain tout patient alors où en sommes-nous en terme de démographie médicale Madame la ministre. Il faut le regarder avec beaucoup d'humilité parce qu'on connaît le constat et les chiffres, mais c'est le moment ou alors qu'on parle d'innovation santé qu'on peut aborder certaines pistes, ce qui serait innovant, Madame la Ministre, ces 2. Comment ça se dire plafonner les installations là où on est sur des territoires surdotées. Pour déverser sur les territoires sous-dotés, je ne cesse de rabâcher là-dessus, mais il existe les moyens réglementaires de le faire avec le conventionnement temporaire sélectif ce qui serait innovant, c'est de permettre aux pharmaciens d'officine de continuer à renouveler systématiquement tout traitement, s'appuyant sur une première prescriptions qui fait état d'Annie agnostique avérée. Ce qui serait innovant, Madame la Ministre, c'est de mobiliser les personnels de santé des armées, j'ai interrogé votre collègue du gouvernement pour savoir qu'ils étaient l'état des personnels, médecins militaires infirmiers pour les utiliser, là où nous sommes en carence, ce qui serait innovant, Madame la Ministre, enfin. Prendre le décret qui est attendu depuis 3 ans je crois, suite notamment à la proposition de la sénatrice Imbert de du Sénat pour déverser les internes en milieu rural, donc il y a des solutions, je ne dis pas que tout a été mal géré dans cette crise, je crois qu'il faut beaucoup d'humilité parce qu'aucun d'entre nous ne s'y attendait, il n'aurait été formé à une telle réponse, mais il y a aujourd'hui des priorités : la santé en fait partie, et donc il faut beaucoup de courage, beaucoup d'audace pour que cette innovation en santé répondent aux priorités qu'attendent les habitants de ce pays, je vous remercie. Merci, cher collègue, enfin, dernier orateur, monsieur Guillaume Chevrollier pour le groupe Les Républicains pour 4 minutes. Merci monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je salue tout d'abord le travail de Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales et d'Annie Delmont Koropoulis Pulis, rapporteur à l'initiative de cette proposition de loi relative à l'innovation en santé santé est issu d'un travail de fond menée en lien également avec notre collègue sénatrice Véronique Guillotin, vous avez en effet présenté en juin dernier un rapport d'information, dressant le bilan du Conseil stratégique des industries de santé 2018 afin de préparer celui de 2021. Le constat que vous faisiez était selon vos mots, celui du déclassement de la France dans le développement et la production de thérapies innovantes en dépit de ses qualités académiques industriels et de recherche, la souveraineté sanitaire de notre pays exige un effort massif pour accompagner le virage des biotechnologies. Il exige aussi une politique de soutien à l'appareil industriel pour favoriser l'émergence de clusters d'envergure internationale, la recherche doit également Rejoindre les standards internationaux en termes de financement, c'est un enjeu capital. La proposition de loi vise notamment à rénover l'évaluation éthique de la recherche en santé, a précisé les objectifs de la politique de recherche et de santé publique à faciliter l'accès aux médicaments et aux traitements innovants et à mieux encadrer l'utilisation des données de santé. Ce texte tend à lever un certain nombre de freins à l'innovation santé et va dans le bon sens, je salue en particulier les dispositions sur l'espace numérique de santé qui doit permettre de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et surtout la coordination des soins qui est fondamental, à la fois pour les patients et également pour faire des économies. Vous revenir sur les articles 21 et 22 textes l'article 21 interdit l'usage des données de santé par les organismes complémentaires à des fins de sélection des risques, la commission a réécrit cet article afin d'éteindre l'application d'une des finalités interdite existant pour l'usage des données du système national des données de santé à l'ensemble des données personnelles de santé je salue cette réécriture, l'article 22 vise à sécuriser le stockage des données en santé, en réservant leur hébergement et leur gestion à des opérateurs relevant exclusivement de la juridiction de l'Union européenne, mais comme l'a rappelé le rapporteur, il n'existe pas encore de solution technique souveraine à même de remplacer Microsoft Azure l'outil auquel la plateforme des données de santé a recouru pour héberger et gérer des données de santé du système national des données alors Monsieur le ministre, dans la discussion générale, tout à l'heure, a rappelé que les données étaient stockées en France mais je rappelle que, dans un avis du 3 février dernier le conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie réclame un appel d'offres pour la plateforme de données de santé, le conseil de la CNAM souhaite qu'un appel d'offres avec la mise en place d'une commission indépendante soit prévue pour choisir un nouvel hébergeur en remplacement de Microsoft pour héberger cette plateforme de donner son avis, qui doit regrouper toutes les données de santé de nos compatriotes, un avis intervient alors que le projet est en suspens depuis fin décembre et que le gouvernement ayant retiré sa demande d'autorisation à la CNIL, indispensable à la pleine mise en Oeuvres de la plateforme, ce repli temporaire justifiée par des motifs techniques mais permettant aussi d'éviter un désaveu sur ce sujet sensible du gouvernement en pleine campagne présidentielle donc le Conseil d'État a reconnu, dans une ordonnance du 13 octobre 2020, l'existence du risque de transfert de données issu de la plateforme données santé vers les États-Unis du fait même de la soumission de Microsoft au droit américain, il y a des gars demandé que des garanties supplémentaires soient mises en place, CNIL, qui partagent cette inquiétude, a estimé que ce risque devait disparaître, donc le ministre Taquet tout à l'heure à relever ce risque en début de discussion générale, donc il nous faut des réponses précises, le gouvernement doit être précis sur le sujet, c'est un enjeu de souveraineté et le Parlement et le Sénat en particulier doit être vigilant sur cette question, je vous remercie.

Qui s'abstient. Il est adopté, jamais on voit l'article 2 qui vote pour. Qui vote contre qui s'abstient, il est adopté. Vous rêvez pas à partir du 3 je vais moins vite à l'article 3 un amendement 27 Madame Pomerol. Oui, merci Monsieur le Président, notre groupe se propose de supprimer l'article 3 puisque notre Phil Condit conducteur concernant l'évaluation éthique des recherches biomédicales et plus particulièrement des cliniques réside des cliniques réside dans l'équilibre entre l'objectif d'une meilleure efficacité et la garantie de l'indépendance des comités de protection des personnes, Pepe pour nous actuellement, cet équilibre est atteint avec la plateforme centralisation de soumission, de ses projets de recherches, l'annuaire des experts pour la montée en compétence concernant les pathologies spécifiques ou la pédiatrie, par exemple, et la possibilité de déléguer certaines recherches du type RIP H3 à des comités d'évaluation éthique de la recherche,

C'est un avis de la commission madame la rapporteure. Merci monsieur le président, les auteurs de l'amendement sont défavorables à la spécialisation CPP et au rattachement des CPLP à des établissements privés, alors que la spécialisation des CPP en pédiatrie en maladies rares et souhaitée par les chercheurs, les encours pédiatres notamment, elle sera utile à la bonne évaluation des projets de recherche dans ces domaines pointus, elle ne remet pas en cause le principe des tirage au sort qui aura toujours lieu certes entre des candidats moins nombreux quant à l'indépendance du CPP, elle n'est pas remise en cause non plus par leur mode d'hébergement, elle est garantie par l'article L. 1123 1 du code de la santé publique et leurs ressources certes insuffisante sont constituées par une dotation de l'État, au reste, la précision à cet article sur le rattachement des CPP ne fait qu'étendre la qu'étendre Il y a déjà des CPP hébergés par des établissements privés par exemple, le centre de lutte contre le cancer, Léon Bérard à Lyon, ils ne sont pas moins un des. Pendant que les autres, pour cette raison : avis défavorable, Bonsoir, monsieur le président, le gouvernement sera favorable à cet amendement il est déjà prévu que les CPP puisse se déclarer compétente ou non en pédiatrie et il y a, il dispose en outre déjà de la faculté de recourir à des à des experts et des spatiale liste en tant que besoin donc pour cette raison, le gouvernement favorable. que nous allons soutenir en effet l'adossement des comités de protection des personnes au centre hospitalier universitaire est une réalité pour la majorité des CPP, l'article 3 propose de le généraliser au nom d'une plus grande efficacité ainsi que pour des raisons de spécialité cependant l'adossement des comités de protection des personnes posent un certain nombre de questions, l'audit de l'Inspection générale des affaires sociales de 2004, a démontré que la garantie de l'indépendance des experts chargés d'évaluer les médicaments reposer essentiellement sur l'existence ou pas de conflit d'intérêts, l'adossement des comités de protection des personnes au sein des structures hospitalières et universitaires, un risque de conflit d'intérêt dans la mesure où les experts, chercheurs, professeurs d'université, les spécialistes cohabiter sous le même toit, si j'ose dire, c'est la raison pour laquelle nous relayons les craintes émises par les associations d'usagers eux- mêmes d'engendrer des conflits d'intérêts en adossant automatiquement des SPP au CHU, faute de pouvoir proposer un modèle alternatif, nous soutiendrons l'amendement 27 du groupe socialiste, je vous remercie. Merci je mais aux voix l'amendement 27 avec un avis défavorable de la commission favorable du gouvernement qui est pour.

Oui, monsieur le président, l'article 5 prévoit de renvoyer à un décret la détermination du rythme des évaluations des comités d'éthique ce renvoi ne semble pas nécessaire, il doit être fixée, je pense, par la loi, c'est tout l'objet de cet amendement, qui fixe un délai de 2 ans suffisamment long pour laisser le temps au comité de produire des résultats suffisamment court pour entretenir la dynamique d'évaluation. Merci, avis de la commission. Merci monsieur le président, cet amendement précise dans la loi que les CPP sont évalués tous les 2 ans, pourquoi 2 ans et surtout pourquoi vouloir figer dans la loi ce qui peut être déterminée souplement par voie réglementaire, donc avis défavorable.

Merci monsieur le président, la procédure donc nous vous sont remplacer quelques mots de situation d'urgence sanitaire, nécessitant la mise en oeuvre sans délai nos recherches par les mots état d'urgence sanitaire défini à l'article L. 31 31 12 la procédure on dérogatoire gérer de désignation de comités d'éthique et de protection des personnes, par le ministère de la Santé, dite Fast Track en dehors donc de tout tirage au sort et directement attentatoire à l'indépendance j'instance, c'est le propre l'on vient de discuter cette procédure exceptionnelle doivent être donc circonscrite au maximum cela dire c'est limiter strictement aux situations d'état d'urgence sanitaire, telle est l'objet, cet amendement, l'argument que le madame la rapporteure nous a opposé au moment de la Commission pour fonder le rejet de cet amendement sur lequel nous aurions perdu beaucoup de trop de temps s'il avait fallu attendre à l'instauration de l'état d'urgence sanitaire pour appliquer la procédure Fast Track aux cliniques dans le cadre la pandémie de Covid 19 n'est pas recevable pour l'avenir, l'état d'urgence sanitaire est désormais inscrit dans le code de la santé publique, ses modalités de mise en Oeuvres largement confie et le Parlement a plus que fait la démonstration, ces 2 dernières années de sa capacité à légiférer dans des délais extrêmement contraint, en situation d'urgence lorsque le gouvernement a décidé ainsi, proposons donc de limiter strictement cette dérogation aux situations d'état d'urgence sanitaire établi. Merci, avis de la commission madame la rapporteure. l'intention des auteurs de l'amendement de bien circonscrire l'hypothèse, des dérogations dues au tirage au sort et de recours à la procédure d'urgence pour soumettre un dossier de recherche ACBB mais je ne crois pas qu'il faille la calqué sur l'état d'urgence sanitaire qui est déclaré par décret en conseil des ministres, pour une raison simple : le temps de l'obtention des connaissances scientifiques n'est pas tout à fait le même que le temps politique, la mention d'une situation d'urgence ou de menaces sanitaires graves nécessitant la mise en oeuvre sans délai d'une recherche semble assez précise, une telle situation peut d'ailleurs précédé la déclaration de l'état d'urgence sanitaire à proprement parler

Qui est contre, il est adopté. à l'article 9 4 amendements en discussion commune le 28 madame Pomerol. Merci monsieur le président, nous souhaitons donc supprimer les alinéas de l'article 9, donc il y a 2 à 8, parce que si nous la faculté pour le comité d'éthique de la recherche de la protection des personnes de déléguer certaines recherches non interventionnelles dites RIP 3 3 un comité d'évaluation d'éthique de la recherche, nous n'estimons pas nécessaire de soumettre les recherches en sciences humaines, portant sur le domaine de la santé à l'évaluation de ces derniers, cela nous paraît même potentiellement dangereux soumettre toute recherche qui serait conduite dans le domaine de la santé et ne visant pas développer les connaissances biologiques ou médicale à l'évaluation préalable d'un comité d'évaluation éthique de la recherche conduit, en effet, du fait de l'étendue des recherches potentiellement concernés à comporter un risque d'atteinte au principe de la liberté de la recherche, c'est pourquoi nous vous proposons de supprimer la création du chapitres du code de la santé publique consacrée aux recherches en santé sciences humaines pour ne conserver que la partie de l'article 9 relatif à la codification des comités d'évaluation éthique de la recherche. Merci Madame Paoli, Gaza, vous allez nous défendre les 3 puisque vous en avez 3 d'affilée 18 19 20. Oui, merci Monsieur le Président, le l'article 9 prévoyait ab initio que les recherches conduites dans le domaine de la santé qui ne visait pas à développer les connaissances biologiques médical pouvait faire l'objet d'une évaluation par le comité de vérification éthique, cette procédure était donc facultative, le texte de la commission l'a rendue obligatoire, cet amendement vise à remettre à l'ordre du jour, ce côté facultatif de la procédure car prévoit une procédure d'évaluation obligatoire va à l'encontre, à notre avis, de l'objectif poursuivi par la proposition de loi savoir simplifier et accélérer les processus de recherche. L'amendement suivant. Porte également sur l'article 9 dont la rédaction initiale ne précisait pas, à l'initiative de qui se déclenchait la procédure d'évaluation le présent amendement vise à préciser que cette procédure se fait à l'initiative du porteur de projet de recherche dernière amendements sur l'article 9, il vise à revenir sur 2 des 4 critères qui sont proposés par cet article sur le 1er critère, à savoir la pertinence scientifique et éthique de la recherche, il ne semble pas pertinent que le comité d'évaluation éthique évalue la qualité scientifique d'un projet de recherche, il est plus pertinent, qui se concentre sur sa compétence, à savoir l'aspect éthique de la recherche, le 3ème critère nous semble aussi contestable et ne nous semble pas pertinent, il consiste à évaluer la qualification du ou des investigateurs, ce n'est pas non plus le rôle du comité que de déterminer quels sont les diplômes ou les expériences qui peuvent autoriser les projets de recherche. Merci, avis du rapporteur de la rapporteure sur les quatre amendements. Merci monsieur le président, alors les 3 premiers amendements.

les 1er amendement supprime la soumission des projets de recherche en santé or loi Jardé au comité d'éthique de la recherche, rebaptisé comité d'évaluation éthique de la recherche, c'est pourtant important et utile, car les recherches or loi Jardé qui nourrissent pour partie les sciences humaines et sociales reste l'angle mort de l'encadrement de la recherche sur la personne humaine, alors que certaines d'entre elles peuvent présenter des risques éthiques pour les personnes par exemple la réutilisation de collections biologiques déjà acquise ou l'utilisation des données médicales déjà collectés à d'autres fins, il est donc important d'encadrer toute recherche réalisée sur l'homme, quelle que soit sa finalité : cela permettra en outre de faire monter les sévères en compétences, ce qui sera profitable à tout le système d'évaluation de la recherche et donc la recherche elle-même dans la pratique académique, la vie d'un suaire et de plus en plus demandés pour publier dans un journal scientifique: la vie restera consultatif et ne portera aucunement atteinte à la liberté de la recherche. Donc les 3 premiers avis défavorable Le 4ème cet amendement allège les modalités d'évaluation de recherche en santé par les CER en supprimant la pertinence scientifique et la qualification de l'investigateur, or ce sont des aspects importants pour assurer la rigueur des recherches impliquant certes pas la personne humaine, au sens de la loi Jardé mais portant néanmoins sur l'homme et sa santé est devant, par conséquent, respecter un certain nombre de prérequis, les critères de pertinence scientifique et la qualification des investigateurs sans qu'il faille interpréter cette notion sont trop strictement semble un minimum. Avis défavorable. Pas pour les mêmes raisons, mais vous savez dans le vote, ça se voit pas, elle avait du gouvernement. Alors avis défavorable sur les 3 premiers, tout comme sur le 4ème j'ajouterai que la capacité d'une d'une recherche à produire des données robustes et valide, apportant un supplément de connaissance par rapport aux connaissances qui existe déjà sur le sujet est une condition du caractère éthiquement acceptable de la recherche en d'autres termes, il n'est pas éthique d'inclure des participants dans une recherche ne produisant pas une de connaissances valide supplémentaires et de plus, la vérification par un tiers de l'aptitude de l'investigateur a réalisé les actes prévue dans le protocole de recherche est indispensable pour garantir, non seulement la qualité des observations et donner de la recherche, mais également la sécurité des participants et donc pour toutes ces raisons, avis défavorable. Très bien, je vais mettre aux voix, successivement, les 4 amendements qui ne sont pas identiques, le 28 2 avis défavorables. Il est retiré. Ah bon. Non, non, président, j'entends bien les arguments qui nous sommes opposés, mais la préoccupation que nous avions dans la suppression de 2 c'est l'alinéa était devancée que par exemple des études en sociologie, on a parlé beaucoup de santé environnementale de l'étude des facteurs extérieurs qui peuvent induire des problèmes de santé si des recherches de sociologie, par exemple, doivent être examinés par 6 comités de recherche, je pense qu'on limite vraiment le rôle de la recherche fondamentale et ça ne nous paraissait j'allais dire à la limite effectivement dangereux pour les maths comme puisqu'on parle là de recherche non à non médical et donc la sociologie par exemple, je ne vois pas pourquoi le seraient incluses dans ces comités de recherche. Merci, allez je vais mettre aux voix quand même l'amendement 28 2 avis défavorables qui est pour.

Oui, monsieur le président, cet amendement est un amendement de suppression de cet article puisque il était évoqué la possibilité de recours au chèque emploi-service pour régler les personnes qui sont dans les CP et on pense que c'est une nous inutile puisque le comité de protection des personnes ne sont pas demandeurs, ils nous ont même dit au cours des auditions qu'ils avaient une très haut aujourd'hui national qui règle et qu'il n'y a plus de problème de paiement et que donc le dispositif ne nous paraît pas viable en l'état, en plus, compte tenu des difficultés d'appliquer des chèques emploi-service qui sont normalement réservés à du travail à domicile pour des personnes qui sont dans les CPE, donc nous proposons de supprimer cet article. qui rend les membres du CVP éligibles à certains dispositifs simplifier l'Urssaf, tels que le chèque emploi service universel, c'était pourtant une proposition de l'IGAS et du Contrôle général économique et financier visant à assouplir les modalités d'indemnisation des membres des comités et les CPP n'y étaient pas hostiles ont simplement fait observer que la création d'un agent comptable unique avait résolu un certain nombre de problèmes, il semble en réalité que le bénéfice du saisis ne puisse pas être étendue aux services publics, ni remplacé par un dispositif analogue, et donc que la rédaction de l'article soit techniquement moins abouti que nous ne le pensions initialement par conséquent avis favorable.

Qui est contre. Il est adopté à l'article 11 Madame Paoli gageant le 21. Oui, merci Monsieur le Président, cet amendement vise en fait à définir les notions de souveraineté, de sécurité, notamment en précisant qu'elles doivent concerner l'ensemble de la chaîne de valeur depuis la recherche fondamentale jusqu'au développement industriel, nous concentrons trop souvent nos efforts de recherche sur la seule recherche fondamentale au détriment des applications industrielles qui sont pourtant essentiels pour la production de médicaments, le développement de vaccins ou la fourniture d'équipements spécialisés. Merci, avis de la commission madame la rapporteure. Merci monsieur le président si je partage les intentions de l'auteur de l'amendement, il me semble déjà satisfait par l'article L 112 1 du code de la recherche, telles que l'article 11 le modifie en effet l'article 11 de la proposition de loi dispose que la recherche publique, vise le renforcement de la sécurité de la souveraineté sanitaire, il va de soi que cela s'applique à la recherche fondamentale qui constituent la majorité de la recherche publique, par ailleurs, dans son état actuel, l'article L 112 1 du code de la recherche dispose déjà que la recherche publique a pour objectif la valorisation des résultats de la recherche au service de la société qui s'appuie sur l'innovation et le transfert de technologies la combinaison de ces 2 dispositions suggère que le développement d'applications industrielles à la recherche fondamentale et déjà l'objectif de la recherche publique. Pour ces raisons, c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Qui est contre. Il est adopté, je mais au voir l'article 23 qui est. Pour. Qui est contre, il est adopté. après l'article 12 Madame Cohen, oui, l'amendement 36. Oui, merci Monsieur le Président, la crise sanitaire, a mis en évidence la mobilisation des établissements publics pour produire en urgence des médicaments critique en appui des actions engagées par ailleurs si d'une part, les ruptures de stocks ont révélé un volet important des dysfonctionnements du marché pharmaceutique nationale, les prix élevés de la thérapie génique, fabriqués industriellement fragilise depuis bien avant la crise sanitaire la soutenabilité de notre système de santé publique, les prix élevés accentue notre dépendance vis-à-vis des firmes des droits exclusifs autour des tables, des thérapies géniques développés ou mise sur le marché, pourtant issu de la recherche financée par des fonds publics, cette dépendance fut de nouveau exposé par le retrait de Blue Bird bio du marché européen au début du mois d'août, après l'échec d'un accord avec les payeurs européen pour le Glaus pardon approuvé pour le traitement de la bêta-thalassémie, c'est une maladie génétique de l'hémoglobine, la base de négociations avancées par l'entreprise pharmaceutique était de 1,8 millions de dollars pour une thérapie à dose unique la production par des structures publiques de thérapies géniques ou cellulaires représente une alternative à cette dépendance vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, la proposition de loi présentée par nos collègues collègues Les Républicains est censé favoriser l'innovation en santé et notamment la recherche dans le domaine de la médecine personnalisée des thérapies cellulaires et géniques ont permis à la médecine personnalisée de faire de grands progrès et représente une véritable innovation et repose sur des informations détaillées concernant l'origine de la maladie de chaque patient avec cet amendement, nous disons chiche autorisant les hôpitaux à produire des produits de thérapies géniques ou cellulaires. oui, on va dire oui, parce que cet amendement vise à préciser que les préparations hospitalières peuvent comporter des produits des thérapies géniques ou cellulaires, l'exclusion de ses produits des domaines des préparations hospitalières ne semble en effet plus vraiment d'actualité, en particulier le développement par certains laboratoires hospitalo-universitaire de médicaments un et comme les quartiers celle qui constitue un véritable espoir dans le traitement de certains cancers du sang aurait du sens pour favoriser l'accès des patients à ces traitements, en dehors même de l'objectif de constitution d'un pôle public de production, le médicament auquel la Commission ne souscrit pas cet amendement peut être utile et nous rappelle le véritable objectif de cette proposition de loi l'accès des patients à des traitements innovants l'avis sera donc favorable. Madame la ministre, non vraiment pas, non je vous sens allez-y. Dans l'avis sera défavorable, c'est même pas chiche, les produits de thérapie génique sont qualifiés de médicaments de thérapie innovante ponctuellement M. TIPP, par conséquent, ces produits ne relèvent pas du régime des préparations hospitalières, les établissements de santé souhaitant produire CM TIPP doivent être autorisés par l'agence de sécurité du médicament et cet encadrement répond aux exigences techniques particulières associées à la production de ces traitements permet d'assurer, surtout au niveau de qualité pour ces médicaments, c'est donc un avis défavorable. Merci madame. Désolé Désolé de votre avis, Madame la Ministre, mais pour notre part, le groupe socialiste et quand j'étais et républicain soutiendra la proposition de cet amendement du groupe CRCE, puisque nous avons d'ailleurs dans le PLFSS introduit cette notion de renforcement des capacités public de production des médicaments, nous avons fait en proposant que la pharmacie centrale des armées ou les déjà glissement de l'AP-HP puisse produire des médicaments ont lieu la crise avait montré que ce combien c'était important au moment du Covid et je crois qu'il nous faut effectivement retrouver une capacité publique de fabrication de ce type de médicaments et éventuellement aussi effectivement des cartes Self, ce qui était évoqué dans l'amendement donc le groupe socialiste soutiendra slogan de dedans. Très bien, elle est jamais aux voix l'amendement 36 donc, avec l'avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est.

Oui Monsieur Président merci cet amendement propose d'ajouter à la notion de médecine personnalisée, celle de télémédecine la télémédecine constitue effectivement un puissant levier pour lutter contre les déserts médicaux, vous le savez tous mes chers collègues et les difficultés d'accès aux soins, il apparaît à cet égard pertinent de permettre à la recherche d'investir ce ce Champ de la télémédecine. S'il avait de la commission madame la rapporteure. Merci monsieur le président, l'extension proposée par cet amendement est assez éloignée de l'objet du texte, par ailleurs, si l'on conçoit aisément que les recherches relatives à la médecine personnalisée, relève bien de la recherche et de l'innovation thérapeutique, c'est plus difficile à concevoir, s'agissant de la télémédecine qui relève davantage de la mise en relation entre les patients et leurs médecins ou bien entre les médecins, au demeurant, les progrès réalisés dans le domaine de la télémédecine au cours des années 2010 suggère que, désormais, c'est la mise en oeuvre concrète d'initiatives qui pose question, bien plus que les recherches et les innovations dans ce domaine, s'il y a donc un enjeu à ce sujet, ce serait davantage celui de la prise en charge des téléconsultations ou du maintien des actes dérogatoires de télé soit créé lors de la crise épidémique qui font d'ailleurs partie des préconisations du Ségur de la santé en ce qui concerne l'intégration à la stratégie nationale de santé d'un volet consacré à la télémédecine cette proposition se situe aux frontières de la recevabilité au titre de l'article 45 de la Constitution, en ce que cette intégration relève des composants sectoriel de la politique de santé publique, pas ne paraît de toute façon pas nécessaire au regard des dispositions déjà existantes sur la télémédecine. Et le thé soins dans le code de la santé publique et de la priorité accordée par le gouvernement à l'accélération du déploiement de la télémédecine

Qu'elles contrent. Il est adopté à l'article 14 2 amendements en discussion commune le 12 d'abord Madame Guillotin. Les tests de dépistage de biologie moléculaire permet en effet aux patients atteints de cancer, de de connaître leur profil génétique et mutationnel et de bénéficier ainsi de thérapies ciblées, mais les médecins rencontrent parfois des difficultés pour récupérer les résultats de ces tests, en raison, notamment, c'est peut-être pas la seule raison de problèmes d'interopérabilité des systèmes d'information, de la même façon, les patients n'y ont que rarement accès, les résultats étant très souvent quasi exclusivement adressé directement au médecin prescripteur dans ces conditions, si le patient a besoin de présenter un jour les résultats de ces tests-là peut s'avérer très compliqué et perturbé le le suivi et les antécédents du patient aussi cet amendement vise à les rendre plus facilement consultables, il est proposé de les transmettre avec l'accord du patient sur son espace numérique santé et c'était l'objet de cet amendement. Et Madame la Sarah d'un amendement proche le 16. Oui, à ses proches, l'objet de cet amendement et de systématiser la transmission des résultats de tests de dépistage de biologie moléculaire aux patients sur son espace numérique de santé de façon à les rendent facilement consultables les patients restent les premiers propriétaires de leurs données de santé quoi qu'il en soit, l'article L-1000 11 13 1 du code de santé publique dispose que le titulaire ou le représentant légal et le seul gestionnaire et utilisateurs de l'espace de santé numérique, il peut donc décidé de proposer un accès temporaire ou permanent à son espace numérique de santé un établissement santé ou un professionnel de santé mais aussi extraire les données de l'espace numérique de santé la possibilité d'inscrire automatiquement les résultats d'un test de sage d'un cancer d'un patient dans MON Espace Santé permettra de garantir un meilleur suivi des patients, telle est l'objet de cet amendement. Oui, merci Monsieur le Président. Les amendements sont très proches, alors donc je vais commencer par l'amendement de Madame. Guyotat cet amendement prévoit l'intégration des résultats de biologie moléculaire dans l'espace numérique de santé, c'est une idée très intéressante, que je salue et qui permettra de garantir un meilleur suivi des patients, mais il y a une demande de retrait au profit de l'amendement numéro 16 de Madame la Sarhane, pour des raisons parce que la

Madame la rapporteure, c'est l'inverse. Avec l'accord, c'est dans le moment où Madame Guillotin, donc si vous voulez la Corse ne comprends pas ce que vous dites là. Non, il y avait de quoi non

et avec plutôt que et me demande de retrait pour l'amendement du même Dieu. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Pour nous, ils sont déjà satisfaits donc. Bon, à l'heure, madame Guillotin, est ce que vous acceptez de retirer votre amendement au profit du 16 de déficit ou le rendre identiques. Comme ça, en fait, 2 amendements, hein, il y a pas de raison donc je considère que le 12 rectifié. Correspond au 16 avec la même rédaction et nous allons, dans ces conditions, avec un avis favorable, si j'ai bien compris de la commission défavorable du gouvernement qui considèrent que ces satisfait le journal Excusez-moi, monsieur le président, mais je souhaitais intervenir avant de dépôt des amendements et j'ai pas lu le droit, c'était assez rapidement, c'était un peu pour souligner, sur le fond le la création de ce forfait de caractérisation de cancer, en particulier en ce qui concerne donc diagnostic génomiques et les biomarqueurs et l'évolution des Worker des bio-marqueurs compagnon, on sait qu'aujourd'hui on a une enveloppe donnée fermé avec en fonction de l'Ondam et certains diagnostics ne peuvent être ensuite fait puisque l'enveloppe a été déjà mangé en cours d'année, et que donc que les hôpitaux sont obligés de se débrouiller comme ils peuvent pour essayer de faire faire ces diagnostics génomiques comme ils le peuvent, je voulais que profiter de la présence de la ministre, vous poser une question justement sur ce sur ce forfait de caractérisation d'un cancer, puisqu'il est dit dans le texte que ce serait sur le budget de l'ARS et j'ai un peu de mal à comprendre comment c'est là l'ARS, qui va fixer ce ce budget, région par région, on a bien répondu en commission, que ce serait identique sur l'ensemble de la France, mais je me demande pourquoi ça n'est pas sûr budget national et c'est pour ça d'ailleurs que ce n'est pas inscrit dans ce texte, c'est puisqu'il faudrait que soit évoquée dans le PLFSS mais j'aurais aimé avoir quand même une réponse de la Ministre sur l'inscription de ce forfait ou est-ce qu'il veut être budgétairement, mais s'il vous plaît. non. Non, bon. Alors je mais on voit donc seulement l'amendement 16 et le 12 qui a été modifiée pour correspondre au 16 avec un avis, je le répète favorables de la commission est défavorable du gouvernement qui considèrent que ces satisfait qui vote. Four. Qui vote contre. Ils sont adoptés. J'ai ensuite un amendement 15 Madame Guillotin.

l'idée du 15 c'est de permettre l'ouverture d'un nouveau forfait en cas de diagnostic de la rechute ou de récidive du 1er cancer et l'Arctique, pardon le l'amendement numéro 14, c'est de proposer que le forfait, donc de caractérisation d'un cancer puissent être utilisés à différents moments du parcours du patient à partir du diagnostic, parce qu'on sait que le le diagnostic qui en fait le besoin de de tests moléculaires peut-être nécessaire d'à plusieurs moments du parcours du patient. Vous avez présenté les 2 très bien avis de la commission sur le XV puis sur le 14 et le gouvernement donnera les 2 avis puis je mettre au vote séparément chacun des 2. Merci monsieur le président, le 15, cet amendement précise que le forfait de diagnostic cancer peut être utilisé en cas de rechute si untel amendement n'a pas été déclarée, c'est qu'il a été interprété comme entrant dans le périmètre du dispositif d'origine, lequel vise tout nouveau cancer il appartiendra alors au texte d'application de préciser qu'une récidive, peut être considéré comme un nouveau cancer. Avis favorable le. 14 cet amendement précise que le forfait cancer Diagnostic cancer peut être utilisé à tout moment dans le parcours du patient, il n'est pas évident qu'une telle précision soit utile, le dispositif de l'article n'impose pas le recours au forfait, à un moment particulier, il appartiendra aux médecins prescripteurs de le déterminer et l'amendement précédent. Le recours au forfait possible civils donc plutôt avis de retrait Madame la Ministre. à l'échelle nationale avec l'INSERM, le plan France médecine génomique alloue un financement annuel dédié au développement de la génomique, en France, tant dans le domaine du soin que dans la recherche par ailleurs dans le cas du plan innovation. Le ministère des solidarités, a d'ores et déjà engagé des travaux sur l'évolution globale du système d'accompagnement des actes de biologie et d'Alain Mathot pathologies innovants afin de permettre de faire diminuer cette pression financière et remettre l'innovation au coeur du dispositif cette approche globale semble plus pertinente qu'un découpage par sous-types d'actes et j'régionalisé. Par ailleurs, pour répondre à votre question madame la sénatrice l'Ondam a déjà une enveloppe sur les tests, il n'y a pas de notion d'ARS et et de fait déjà accès pas d'enveloppe supplémentaire en fait c'est déjà acceptée par principe voilà. Bien madame Guillotin, vous maintenez les 2. Le 14, d'accord, donc je vais mettre aux voix l'amendement 15 avec un avis favorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement qui est pour le 15. Qui est contre. Il est adopté et le 14 n'est pas soumis au vote je mais aux voix, l'article 14 ainsi modifiées qui est. Qui est contre, il est adopté, jamais on voit l'article 15 qui est pour. Qui est contre. Il est adopté, après l'article 15 un amendement si Monsieur Milon. Oui, merci Monsieur le Président, cet amendement fait vise à confier à la Haute autorité de santé une mission visant à dresser un inventaire des mécanismes d'accès précoce en France pour les produits de santé innovant, ce recensement pourrait donner lieu à une évaluation annuelle dans modalités d'utilisation en collaboration bien sûr avec l'Agence de l'innovation en santé, dont la création a été annoncée par le plan Innovation 2030, présenté en juillet 2021 enfin, le président de la République, cette nouvelle mission de la Haute autorité de santé contribuerait à pallier le manque d'informations disponibles relatives à la prise en charge des produits innovants permettrait également de garantir un suivi annuel de efficience des mécanismes de diffusion de l'innovation en santé.

celle de faire un état des lieux des mécanismes d'accès dérogatoire et temporaire pour les produits de santé innovant et de proposer des mesures de simplification, une telle mission nouvelle n'apparaît pas utile les dispositif d'accès à l'innovation sont bien connus des industriels et la communication sur les différents dispositifs c'est encore employé en ligne depuis la crise sanitaire c'est encore déployés en ligne depuis la crise sanitaire, en outre, la HAS organise déjà des rencontres d'orientation stratégique des rencontres précoce et des rendez-vous près des pots qui permettent d'informer, d'orienter au mieux les industriels pour rendre lisible la cartographie des différents dispositifs, la réforme de l'accès précoce de juillet dernier, a déjà permis d'unifier et simplifier et accélérer les dispositifs d'accès dérogatoire aux médicaments depuis moins d'un an, le bilan à 6 mois et positif en termes de délais et de dispositifs évalué le forfait innovation a été profondément revu et simplifié en 2019, 2020 et un dispositif complémentaire d'accès transitoire pour des dispositifs médicaux a été créé en 2021 en outre des rapports et bilan sont déjà prévues par la loi concernant la réforme de l'accès précoce et la HAS va publier bientôt de tels bilan annuel dans ses rapports d'activités prévues par la loi. Donc c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre, avis défavorable. Qu'il est maintenu, il est retiré, il est retiré. à l'article 16 monsieur dessus. merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est une prise de parole pour vous alerter sur cet article 16 qui a été pointée du doigt aujourd'hui même par l'Observatoire pour la transparence des médicaments comme comprenant une mesure introduite à l'heure à la demande du lobby des entreprises du médicament principalement donc les multinationales du secteur, il s'agit de fixer le prix des nouveautés thérapeutiques pour lequel les données cliniques seraient encore insuffisante par un nouveau critère la valeur thérapeutique relative, vous l'aurez compris, tout est dans le relatif et le flou de ce que sa disposition introduit, il est à redouter que soit ainsi renforcer le déséquilibre entre le régulateur public le comité économique des produits de santé et les firmes celles-ci auront encore plus de pouvoir pour entamer les négociations avec un prix exorbitant, alors même que le produit ne serait pas pleinement évaluer s'il en était besoin, la crise sanitaire à l'acte de laquelle nous peinons à sortir, a mis en exergue le besoin de transparence, de nos concitoyens vis-à-vis des médicaments, et particulièrement de la manière dont leurs prix sont fixés cette transparence démocratiquement vital est également indispensable à l'adhésion de nos concitoyens aux politiques sanitaire, y compris en temps de crise aussi pour répondre à ce besoin de transparence, notre groupe écologiste a déposé des amendements suivants d'évaluation pour les caisses sur lesquels s'appuie le comité économique des produits de santé, les investissements réels au titre de la recherche et développement du financement public et de la recherche, et d'autre part à rendre publiques les données permettant de réévaluer périodiquement les valeurs thérapeutiques relatives des médicaments, en espérant que notre haute assemblée sera avancée vers plus de transparence, notre groupe défendra donc ces propositions, je vous remercie. Oui, merci Monsieur le Président, l'article 16, propose de modifier les critères de fixation des prix, en ayant recours à la notion de valeur thérapeutique relative ce mécanisme existe déjà sous l'appellation contrats de performance mais n'a été que peu utilisée en raison d'ailleurs du faible intérêt de ce dispositif, surtout, ce mécanisme a été décrié par la Cour des comptes, qui dressait un bilan plutôt accablant 2017, je cite, dans la quasi-totalité des cas l'hypothèse favorable associé aux contrats de performance, c'est-à-dire la démonstration en vie réelle d'une efficacité supérieure du produit ne s'est pas vérifiée pour les associations d'usagers, ces contrats renforce le déséquilibre entre les industriels et l'assurance maladie qui est contrainte comme nous l'avons déjà souligné, d'accepter des tarifs très élevés, sans possibilité d'évaluer les dispositifs qui ne concernent qu'un faible nombre de malades et donc rend impossible une renégociation vers le bas de ces mêmes tarifs pour ne prendre qu'un exemple, un traitement par exemple, c'est le cas de le dire, contre l'hépatite C a été facturé 40000 euros l'unité à l'assurance maladie, alors que que son coût de production se situait autour de 265 euros, comme je l'ai souligné dans la discussion générale, il est vraiment urgent de retrouver une maîtrise publique dans la politique du médicament, l'opacité et le manque de traçabilité de ce mécanisme est tout à fait inacceptable et d'autant plus que vous savez pertinemment, mes chers collègues, que ces innovations dépendent en réalité d'un financement public dans l'ensemble de la chaîne de l'innovation pharmaceutique de la recherche fondamentale à la production c'est pour ces raisons que nous demandons la suppression de l'article 16. Merci monsieur le président, c'est un avis défavorable à la suppression de l'article 16 qui propose un nouveau mécanisme d'accès au marché des médicaments innovants l'hypothèse visée et celle des médicaments destinés à Detroit de cohortes de patients atteints par exemple de maladies rares, ce n'était pas le cas de l'hépatite C n'est pas une petite cohorte, comme le relevait déjà le rapport de notre collègue Jocelyne Guidez sur la proposition de loi relative aux cancers pédiatriques au regard de leur caractère particulièrement innovant et de l'étroitesse des populations concernées pour chaque pathologie l'efficacité de certaines molécules développées spécifiquement dans le traitement des cancers pédiatriques ne peut bien souvent être étayé par des études cliniques suffisamment large, d'autant qu'il s'agit généralement de traitement de dernière intention qui emprunte des mécanismes d'action en rupture avec les thérapies

d'où le mécanisme proposé à l'article 16 qui propose d'asseoir sur un nouvel indicateur la fixation du prix du médicament, il peut sans doute être améliorée, mais il maintient ouvert à débat nécessaire sur la tarification des médicaments innovants. L'avis du Gouvernement est favorable sur cet amendement, nous sommes favorables à cet amendement pour 2 principales raisons : d'abord, les laboratoires sont responsables de leur plan de développement et peuvent bénéficier de rencontre précoce avec l'ANSM et la HAS, ils ont en outre la possibilité d'avoir accès au marché, plus de 2 ans avant l'autorisation de mise sur le marché, l'accès aux patients est assurée, avec une prise en charge, un recueil de données est alors mis en place en vue de l'évaluation de droit commun et, enfin, il est particulièrement complexe d'envisager une inscription dans le panier de soins remboursables ou d'espérer un accord conventionnel lorsque les données ne permettent pas d'étayer la valeur du produit, donc favorable. Bien, je vais mettre aux voix l'amendement 41 avec un avis défavorable de la commission favorable du gouvernement qui est pour.

monsieur le président, un nombre croissant de médicaments représentant des innovations de rupture obtiennent une autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament sur la base de données incomplètes du fait de leur enregistrement précoce ou de données qui par nature ne pourront être obtenus qu'vie réelle après la commercialisation du produit ses médicaments ouvrent des perspectives d'efficacité hors du commun qui doivent être confirmés par l'obtention de données complémentaires à une date ultérieure ayant obtenu une AMM, il dispose de données démontrant une balance bénéfice risques favorable, or lors de l'évaluation de l'amélioration du service médical rendu la HS se prononce ce strictement sur les données constater et s'interdit la possibilité d'anticiper l'obtention de données futur en conséquence les médicaments concernés obtiennent un niveau d'SMR dégradé qui est révisé à l'obtention des données définitives ce processus en 2 temps, crée des difficultés d'accès au traitement, les négociations de prix et l'inscription sur la liste en Suisse notamment, se heurtant à laisser initial dégradé qui ne reflète pas le réel potentiel du produit, la mise en place d'une AS maire conditionnel qui autoriserait la HAS a anticipé l'obtention des données futur permettrait de résoudre la problématique de ces médicaments a données incomplètes, de l'expérimentation proposée dans l'article législative du code de la Sécurité sociale portant sur la négociation de prix peut porter à confusion quant à l'objectif et au périmètre de l'expérimentation, il apparaît plus pertinent de ne pas codifié cet article et de préciser le périmètre et les modalités de les vols de l'évaluation concernés.

la notion de valeur thérapeutique relative est utilisé depuis le CSIS 2013 pour désigner un nouvel indicateur unique agrégeant le SMR qui détermine l'accès au remboursement et l'qui détermine le prix, elle a fait l'objet de propositions en ce sens de 2 rapporteurs généraux successifs du budget de la Sécurité sociale au Sénat en 2013 et 2014 la notion a été reprise par Dominique Paul-t-on dans un rapport de novembre 2015, puis dans le rapport de Gilbert Barbier et Yves Daudigny, de joie, de juin 2016 dans celui de Catherine Deroche, Yves Daudigny et Véronique Guillotat de 2018 et régulièrement depuis, l'intérêt pour cette notion repose sur l'idée qu'un nouveau système d'évaluation est nécessaire, en particulier pour les médicaments très innovants pour lesquels, par hypothèse, l'étroitesse de la population cible et le caractère nouveau du mécanisme rend toute comparaison difficile avec le à un médicament existant, la notion de VTM semblent donc plus appropriées que celle d'un SMR, la détermination de cette GT-R ne sera certes pas évidente, les travaux et réflexions de la HAS fournissait toutefois quelques pistes qui insistait sur la quantité d'effets tant en termes d'efficacité, de qualité de vie et c'est important que de tolérance et eu égard à la gravité de la maladie, la pertinence de l'effet, la qualité de la démonstration la place dans la stratégie thérapeutique sans doute peut-on encore affiner cette base d'analyse

Oui, monsieur le président, ainsi le délai maximal de révision qui est fixée par cet article semble raisonnable pour actualiser régulièrement le prix au plus juste il nous sommes que la durée totale de l'expérimentation est insuffisante huit guerre en période de retour sur investissement pour le développement de médicaments vraiment plus innovant, c'est pourquoi le présent amendement vise à allonger la durée maximale de l'expérimentation de 5 à 10 ans. Merci monsieur le président, cet amendement étant à 10 ans au lieu de 5 la durée de l'expérimentation proposée à cet article : la durée de 5 ans semble suffisante pour obtenir un 1er aperçu de l'intérêt du dispositif : avis défavorable. Du gouvernement

Merci monsieur le président, donc c'est un moment qui vise à assurer la transparence des prix du du médicament qui est un enjeu majeur de démocratie sanitaire qui devrait être l'objectif de tout public de santé, puisque c'est l'objectif de s'assurer de l'accès de toutes et tous à la santé, or depuis 2005 le prix des médicaments innovants a augmenté de 200 % ces prix croissant ne pèse pas uniquement sur les patients mais également sur les dépenses de l'assurance de l'assurance maladie, nos concitoyens doivent alors pouvoir connaître la contribution du financement public dans le développement par les entreprises de traitement privé il apparaît notamment que la participation publique n'a eu aucune influence sur le prix des médicaments qui devrait pourtant être revu à la baisse, en conséquence, des associations comme Aides ont cherché par des campagnes comme Alerte médicament a attiré l'attention des pouvoirs publics sur les enjeux d'une transparence des prix, notamment pour les traitements contre le VIH ou les hépatites, c'est pourquoi nous proposons par cet amendement d'ajouter les investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de la recherche au critère de fixation du prix des médicaments sur lesquels s'appuie le communiqué le comité économique, de produits de santé, c'est le PS, pour la même durée expérimentale de 5 ans prévu par cet article, je vous remercie. Merci le 29 madame Pommier. Merci monsieur le président, c'est notre amendement 29 dans le même sens que celui qui vient d'être présentée puisque introduire un critère de valeur thérapeutique relatif dans la fixation du prix des médicaments dits innovants est une demande récurrente en fait de l'industrie biomédicale et du même en particulier et la majorité sénatoriale cherche depuis de nombreuses années à satisfaire cette demande du il convient quand même à tout le moins, dans le cadre de l'expérimentation de 5 ans qui est ainsi proposé, et ce d'autant plus que toutes les données ne seront pas disponibles pour apprécier et l'efficacité et la sécurité de ces 2 médicaments, le définir, cadre de fixation des prix le plus équilibré possible entre la valorisation pour l'industriel et la charge financière pour les comptes de la Sécurité sociale, actuellement dans la fixation des prix, les investissements qui sont réalisés par les industriels, notamment en recherche et développement et en production peuvent être prises en compte dans la définition du prix, selon l'article 18 de la record Khadr du 31 12 2015 entre CNPF et le l'M mais inversement, l'État lui ne veut pas prendre en compte les investissements en R et D, Directs ou indirects qui va effectuer pour fixer le prix d'un médicament, le cas de fixation des prix donc déséquilibré au bénéfice de l'industrie pharmaceutique et et au détriment des comptes publics et de la protection sociale, notre amendement vise donc, comme le président introduire des critères de fixation d'un prix juste, à savoir les coûts réels de production, c'est en plus par rapport au précédent et les investissements publics en RD dans le quart d'une expérimentation, sollicitée par l'industrie du médicament elles-mêmes. Avis de la commission sur ces deux amendements madame la rapporteure. d'une telle information pour jouer son rôle qui lui est communiqué par les industriels, sur le fondement de l'article L 162 17 4 3 du code de la santé publique sur le fond, la seule connaissance de cette information est très difficile à obtenir comment obtenir d'entreprises mondiales, montant du financement public perçu surtout partout par leurs filiales et comment définir ces Liens public la générosité par exemple par le biais du Téléthon est-elle considérée comme du financement public, comment prendre en compte les rachats successifs d'innovation et une fois l'information obtenue comment exactement pondéré dans le prix du médicament, la part de financement public et privé, donc l'avis sera défavorable à ce stade. Sur les 2 on est bien d'accord hein madame la rapporteure très bien avis du gouvernement. Même avis sur les 2 le le niveau d'investissement public en recherche et développement, où les coûts de production ne présage en rien de l'intérêt clinique du médicament développé si tenté que les recherches aboutissent à la mise sur le marché du 10 médicament cette proposition pourrait donc s'avérer contre-productive et conduire à accroître les dépenses à l'assurance maladie pour des médicaments ayant eu des coups de RND élevé mais sans valeur thérapeutique démontré : avis défavorable, donc sans compter qu'un telle critères risquerait in fine et d'inciter les hommes, les industriels à réaliser une recherche de moins bonne qualité, quitte à en faire quantité vous quantitativement plus j'arrive pas le dire ou à ne pas travailler à la maîtrise de leurs coûts de production, je mets de l'animation. Donc, avis défavorable sur les 2, je vais mettre aux voix successivement le 32 et le 29 avec 2 avis défavorables dans les 2 cas, 32 qui est.

Roche. Le président : permettre à la Haute autorité de santé, de faire des études sur la valeur thérapeutique, des médicaments et c'est une avancée dont nous devrions tous nous féliciter dont nous fait ici félicitant nous en tant qu'écologistes, c'est une revendication de l'orgue date des acteurs de la santé que de pouvoir faire des essais comparatifs avec les meilleurs traitements disponibles, la réévaluation périodique est également une mesure positive toutefois l'enjeu majeur et la qualité des bases de données sur lesquelles s'appuie l'expertise de la Haute autorité de santé rendre ces données publiques nous paraît pour le moins essentiel, voire nécessaire, cela permettrait de faciliter les contre-expertise d'acteurs indépendants comme la revue médicale Prescrire dont je tiens à souligner et à saluer ici le travail, la transparence des bases de données permet alors de renforcer la confiance de nos concitoyens dans ces traitements innovants et de faciliter le travail journalistique et scientifique de contre-expertise de la société civile, en conséquence, cet amendement attribue à la Haute autorité de santé la tâche de rendre publics les 10. Merci monsieur le président, cet amendement prévoit de rendre publiques les données santé envie réelles Servent à réévaluer périodiquement la valeur thérapeutique relative cite : renforcer la confiance des patients dans ces médicaments et, d'autre part de faciliter le travail journalistique et scientifique de contre-expertise de la société civile, on peut douter d'une part que la défiance a priori à l'égard de la Haute autorité de santé soit de nature à renforcer la confiance des patients et, d'autre part qu'il faille confiée à la société civile, la contre-expertise toutes les expertises, mieux vaut sans doute se concentrer sur les moyens de permettre aux experts d'exercer leur mission dans les meilleures conditions, donc avis défavorable. Avait des gouvernements même avis.

Merci monsieur le président, cet amendement vise à diversifier la composition du comité économique des produits de santé, le CPS, en y intégrant ce qu'on appelle des acteurs de la société civile organisée, à savoir des personnes impliquées dans ces des associations et ONG qui travaillent sur les enjeux de santé le CNPS et l'organisme interministériel chargé de fixer le prix d'un médicament, toujours dans une logique de démocratie sanitaire, il est essentiel d'y intégrer des personnalités qualifiées de la société civile impliqués dans ces associations et ONG, spécialiste du sujet des associations comme Aides, Médecins du Monde ou prescrire pourrait en effet relayer les préoccupations citoyennes relatives aux prix des médicaments est complété expertise institutionnel ce soutien permettra ainsi de renforcer la démocratie sanitaire pour éviter tout risque de conflit d'intérêt, ces personnalités qualifiées devront être indépendantes, c'est-à-dire dénué de tout lien avec des entreprises et l'abattoir pharmaceutique l'objet de cet amendement, merci. Merci à avis de la rapporteure. Merci monsieur le président, cet amendement précise qu'un collège de personnalités qualifiées, participe aux travaux du CNPS, le temps de l'expérimentation prévue à l'article 16 l'amendement ne précise pas comment ce collège serait intégrée à la composition du GPS ni dans quelle mesure il participe aux décisions relatives à la fixation du prix des médicaments, on comprend bien à nouveau l'intention qu'on consistant à faire la transparence sur l'activité des autorités de régulation une fixation des prix mais le le dispositif ne semble pas très aboutie, mieux vaudrait s'efforcer de donner à ces instances les moyens d'exercer sereinement leur mission, sujet sur lequel nous pourrions en effet revenir quelques jours la PrEP proposition de loi n'ambitionnait pas de rénover l'ensemble du système d'évaluation et de tarification des médicaments avis défavorable. Avis du Gouvernement défavorable. D'accord. Je mais on voit le 35 avec 2 avis défavorables qui est.

dès le PLFSS 2018 et qui avait été source de discussions qui sont restés nous abouti jusqu'à présent, et ça me paraît tout à fait important parce que c'est vraiment une méthode innovante qui propose une nouvelle, une utilisation testimoniale éclairée surveillée, ça s'adresse surtout à ceux qui ont des troubles cognitifs et vous savez que la recherche dans le domaine est particulière, ça nécessite énormément de temps entre le moment où il y a des découvertes qui sont faites avec une amélioration des découvertes qui se retrouvent sur la paillasse des laboratoires et qui mettent 15 ans avant de se retrouver sur l'étagère des pharmaciens en conséquence, je vous propose le le droit à essayer, comme il existe ailleurs, il a été votée récemment aux États-Unis, c'est-à-dire nisation testimonial éclairé surveillée c'est elle suppose que l'implication et la responsabilité du malade qui souhaite par instinct de survie, prendre le risque d'améliorer son état de santé grâce à des médicaments qui en ont pas encore suffisamment prouvé leur efficacité, l'existence d'un risque différencie cette utilisation testimonial de l'usage compassionnel du médicament c'est une une utilisation bien sûr éclairer puisque elle découlerait véritablement d'un choix du malade qui doit être conscient des risques qu'il encourt, elle doit être enfin surveiller parce que c'est la vie du patient qui est en jeu, voilà l'objet de cet amendement. Merci monsieur le président, cet amendement crée un nouveau mode d'accès aux médicaments en phase d'essais cliniques pour les personnes atteintes de pathologies graves dégénérative hein tels mécanismes est d'abord une proposition d'espoir d'amélioration pour les personnes privées de solutions thérapeutiques, l'utilisation du médicament semble suffisamment encadré puisque dépendant d'hypothèses sur demande du patient et de manière surveillée à l'opposé de ce qui nous est proposé ici en ce moment, on a à notre époque, Ueli l'idée du suicide assisté ou de l'euthanasier reçoit un soutien donc il serait curieux maintenant de Niamey Fuster davantage de suspicion à l'égard d'une procédure vit une vent visant non pas à abréger la vie, mais à la prolonger, à la demande du malade, j'observe enfin que le Sénat avait voté un amendement presque identique lors de l'examen du Plfss pour 2018, donc avis favorable. Madame la ministre. coût du Gouvernement est défavorable, la réglementation relative aux recherches impliquant la personne humaine est une réglementation protectrice des personnes qui participent à des recherches pour des raisons évidentes d'éthique en effet la recherche n'est pas le soin et réaliser des à. Intervention médicale non parfaitement justifiée doit répondre à des fortes exigences éthiques, le gouvernement est défavorable à votre amendement car le dispositif qu'il porte, ne semble pas répondre à un besoin non couverts par les accès compassionnel nominatif ni suffisamment encadré sur le plan de la sécurité ou sur le plan éthique. Merci bon oui, monsieur, non, non, l'auteur de l'amendement d'abord aller à vous monsieur le oui. Vous le retirez vous le maintenez. Du calme alors c'est lui qui va parler, allez, on n'est pas la parole à sa place. Merci,

Parce que ce sont des millions de personnes qui sont concernées par les troupes cognitifs, on n'arrive pas à trouver des molécules innovantes et pourtant, on sait qu'elles existent, simplement c'est très compliqué d'les maths derrière sur le marché, c'est la raison pour laquelle il me paraît important, comme ça se fait dans d'autres pays, de trouver une voie nouvelle, ça concerne quand même des millions de personnes, quoi, et on les laisse tranquillement sans efforts, on les laisse au fil du temps dans un état de santé qui se dégrade et qui coûtent très cher à la société, c'est la raison pour laquelle les et les personnes qui souhaitent bénéficier d'un protocole particulier par l'instinct de survie, elle souhaite essayer, c'est l'utilisation tétines de Montréal je souhaite essayer ce médicament là ça servira à d'autres et puis ça permettra peut-être d'améliorer mon état de santé, mais surtout c'est une une action particulièrement éthique puisqu'elle consiste à prendre le risque à disposition, celui de la recherche pour le mettre effectivement au service d'autres personnes, c'est la raison pour laquelle il me sens mes chers collègues, qu'il faut aller vers cette voie nouvelle qu'effectivement il ne voient particulière qui existent d'entres autres pays qui est reconnu également sur le plan Euro que PAI, qui permettrait, me semble-t-il, de répondre à l'attente d'un certain nombre de patients. Fournir. Merci monsieur le président, nous comprenons bien la question qui se posait par par Monsieur Savary et effectivement les difficultés qu'on est les 4 conditions difficiles qui se présente au au médecin, quand on a des patients sur le corps pour lesquels on n'a rien à proposer d'existant et effectivement laissé de nouvelles molécules, pourrait être une solution mais il me semble avoir compris moi ou j'ai certainement, de mal compris, mais que l'objectif de ce qu'on a mis dans l'accès précoce pour les patients n'aime pas ces thérapeutiques déjà sur le PLFSS 2021 et l'accès Direct, cet homme né en 2022 aller dans ce sens-là, et on n'a pas encore l'expertise sur ce donne l'accès précoce et ce que va donner l'accès Direct comme propose encore une institution et je crois que Monsieur 1000, on parlait tout à l'heure de 2000 feuilles qu'il faudrait faire un bilan de mille-feuilles, me suis non je voulais justement pour une fois soutenir votre votre amendement pour qu'on y voit clair dans ce mille-feuilles là et je trouve que là, on a encore un processus qui viennent complexifier la compréhension de ces différentes accès compréhension qui est déjà difficile.

chaque année, à chaque Plfss, nous avons la même réponse : le problème c'est pas, c'est pas les médicaments innovants en tant que telle, le problème c'est les patients qui arrivent en fin de soins habituels, y compris certains types de médicaments innovants autorisé et qu'on sait que, il y a plus rien à faire d'autre que d'essayer quelque chose qui n'est pas encore complètement établies au niveau de la recherche humaine, c'est ça, avec évidemment l'accord ou du patient ou l'accord de la famille, c'est ce que propose aux Rennais Paul Savary depuis pas mal de temps et je pense que nous n'avons pas le droit aujourd'hui de refuser cette chance, nous n'avons pas le droit de donner une perte de chances supplémentaire à quelqu'un qui, de toute façon, est arrivé à la fin de tout ce qu'on pouvait faire, y compris dans les et dans les médicaments innovants, c'est donc c'est le but de l'amendement de de pas. Un jeu mais aux voix l'amendement, hein, avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour.

d'innovation peu pionnière c'est un amendement propose la mise en place d'un budget décentralisée dédiée aux équipes pionnières, ce budget sera strictement fléchés auprès des équipes hospitalières pionnière de référence est octroyée en contrepartie d'une collecte et du partage des données préliminaires quant à l'utilisation du dispositif médical innovant et de l'acte qui est associé, on parle bien maintenant de dispositifs médicaux, l'accès à un dispositif médical innovant pour un patient et un professionnel de santé est théoriquement possible, possible, dès que le marquage CE est obtenu ça mais sa prise en charge par l'assurance maladie n'intervient toutefois qu'après évaluation de la Haute autorité de santé et inscription sur la LPPR ou au financement dans le cas de GHM or d'une part, les délais d'évaluation et d'inscriptions ne sont pas compatibles avec l'accès précoce aux innovations pionnières, d'autre part une méthodologie d'évaluation sont difficiles à satisfaire un stade d'usage précoce d'un dispositif et restent souvent inadaptées au contexte particulier d'émergence d'une innovation, je vais m'arrêter là parce que je serais trop long, je voudrais juste dire que les dispositifs médicaux, ça n'est pas seulement un pansement ou un plâtre, ça peut être aussi une valve cardiaque et là l'urgence existe. Alors cet amendement propose de faire financer par l'enveloppe des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, c'est-à-dire des dispositifs médicaux innovants, or il existe déjà le forfait innovation qui permet déjà des prises en charge dérogatoire et de dispositifs médicaux innovants. Ces derniers doivent disposer de données établissant que son utilisation est susceptible d'apporter un bénéfice important pour la santé ou de réduire les dépenses de santé, la prise en charge dérogatoire est conditionnée par la mise en place d'une étude clinique par le demandeur afin de confirmer le bénéfice important de cette nouvelle technologie pour la santé, le forfait innovation est accordée par les ministres chargés de la santé et la sécurité sociale, après avis de la HAS, ce dispositif a d'ailleurs été largement simplifié et rénové en 2019, 2020 par ailleurs, il existe un certain nombre de programmes de recherche hospitaliers destiné à sécuriser à cadrer la l'accès à l'innovation, le programme de recherche sur la performance du système de soins, programme de recherches médico-économique et programme hospitalier de recherche clinique, donc ce sera un avis défavorable.

Oui monsieur le en commission un amendement de la rapporteure à conditionner l'accès au système national des données de santé à la validation du protocole de recherche par le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé cette condition : ne pas restreindre l'ouverture du SDS en alourdissant les procédures administratives d'accès, elle nous semble ainsi nuire à l'objectif même poursuivi par le SNPL. Alors avis défavorable, l'amendement vise à supprimer les conditions d'accès ou FNDS prévue par l'article 20 pour évaluer les traitements vie réelle, si les industriels doivent déjà remplir des conditions particulières liées au régime de protection des données personnelles, il n'existe pas des dispositions juridiques tangible visant à obtenir un retour de la part des industriels, à la suite de la l'accès ou FNDS, ou à s'assurer de la validité scientifique de la recherche menée, c'est précisément ce que vise l'article 20 l'évaluation en vie réelle des traitements par les industriels, doit faire l'objet d'une étude remise à l'ANSM et d'une validation des protocoles de recherche en résumé, on ne saurait autoriser l'accès à une base de données aussi précieuse que le SDS dans sans ces garanties et contreparties minimal qui vont dans le sens de l'application du principe de transparence, corollaire du plein déploiement des potentiels des données du SDS pour favoriser les recherches sur les traitements innovants. Ce sera donc encore une fois, une demande de retrait ou à des fois un avis défavorable. La ministre. Avis défavorable ah oui. Et ça. Madame Paoli, il est retiré, ils retiennent 2 amendements identiques, le 3 Madame Lassaad. Merci monsieur le président, en 2019 la loi relative à l'organisation de transformation du système de santé a permis la création de la Health Data le décret 2021 848 du 29 juin 2021 relative au traitement des données à caractère personnel dénommé système national des données de santé prévoit les modalités de gouvernance et de fonctionnement du système national des données de santé dans le périmètre est étendue à de nouvelles bases de données, il permet ainsi au Health Data hub d'être coresponsables du traitement du système national des données de santé au même titre que la Caisse nationale d'assurance maladie, structure publique, le Health Data hub ambitionne d'accompagner des porteurs de projets, en leur permettant d'accéder à des données de santé pour trouver les solutions améliorant la santé des personnes ces données proviennent notamment du système national des données de santé majoritairement de sa base principale rassemblant les données issues de l'assurance maladie, données de prise en charge de soins codage détaillé des médicaments délivrés des actes techniques des médecins consultation médicale, paramédicale, dispositifs médicaux prélèvements biologiques, elles proviennent également des établissements de santé ou encore de santé publique France la création de cet outil prometteur a été saluée par les acteurs du système de santé qui rappelle également je concernant la constitution des bases de données, leur renouvellement, afin de permettre l'optimisation des projets de recherche, les chercheurs recommandent de mettre à jour régulièrement les bases de données pour disposer de données à jour ces données actualisées permettront de mieux rendre compte de l'état de santé des Français et de leurs besoins médicaux, par conséquent, l'amendement propose de mettre à jour trimestriellement et non plus annuellement la base principale du système national de santé. Merci madame Guillotin même amendement défendu avis de la commission sur 7, ces 2 amendements identiques. Merci monsieur le président, les amendements 3 13 sont identiques et vise à demander à la plateforme des données de santé de mettre à jour trimestriellement les données du DS l'avis sera défavorable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, dans la mesure où il vise à assurer la mise en oeuvre concrète des missions qu'il assigne au et CNDS il constitue une disposition réglementaire et non pas la référence au décret du 29 juin 2021 comprise dans l'objet confirme s'il en a été besoin que la loi n'est pas le lieu adéquat pour introduire une telle disposition sur le fond, pour ce qui concerne la base principale du FNDS l'amendement serait ou bien inutile ou bien vraisemblablement contreproductif les données ambulatoires font l'objet déjà des mises à jour mensuelle il n'apparaît dès lors pas utile de proposer une mise à jour trimestrielle les données hospitalières font également l'objet de les remonter mensuelle donnant lieu à une version consolidé annuel qui permet d'ajuster progressivement les données des mois précédents, pourra l'améliorer la qualité, la référence est annuel, pour des raisons de qualité et de fiabilité des données, en effet, si la période de référence était le trimestre on observerait des variations trop importantes d'un trimestre à l'autre du à des effets de rattrapage ce qui entamerait fortement la fiabilité des données et leur intérêt pour le chercheur, toutefois, grâce au dispositif de Fast Track mises en oeuvre depuis la crise sanitaire, si un chercheur souhaite effectuer une étude sur des données trimestrielles, il peut le faire, elles seront simplement de moindre qualité que les données annuels consolidés pour toutes ces raisons, l'avis sera donc défavorable pour les 2. C'est,

Mais aux voix, l'article 20 qui est pour. Qui est contre est adopté je mais au moins, l'article 21 qui est. Pour. Qui est contre, il est adopté à l'article 22 l'amendement 26 Madame Paoli. Oui, monsieur le président, ce sera une ultime tentative pour ma part, un amendement qui vise à renforcer la mesure qui est proposée, relativement à l'hébergement et la gestion des données en y intégrant aussi la notion de protection des données dans la liste des prérogatives attribuées à des acteurs européens, c'est un ajout qui peut paraître anodin, mais qui a pour double Avantage de garantir la maîtrise du stockage des données de bout en bout, et de favoriser le développement d'acteur européen de la cybersécurité en santé, la protection des données, mes chers collègues, ça me semble assez important. Merci, avis de la commission. Madame Paoli, je suis désolé. Avis défavorable, en effet, l'article 22 vise à tirer les conséquences de plusieurs avis de la CNIL, pris à la suite de l'arrêt serait mieux de juillet 2020, qui avait remis en cause l'accord Privacy Shield conclu avec les États-Unis au motif que le caractère extra- territorial de la législation américaine ne permettait pas de garantir un niveau de protection des données de citoyens européens équivalent à celui assuré par le règlement général sur la protection des données, il réserve ainsi un opérateur placés sous juridiction de de l'Union européenne, l'hébergement et la gestion des données du FNDS DS dans la mesure même où il sera placé sous juridiction européenne l'obtient l'opérateur verra sa politique de gestion des données soumises au RGPD qui offre les garanties de protection parmi les plus élevés au monde, l'article 22 remplie donc l'objectif visé par amendement qui est dès lors sans objet.

Ah ben il fallait lever la main, Madame Cohen vous savez c'est c'est comme partout, et c'est pour ça que j'ai attendu un moment. Bon, vous voulez une explication de vote ne vous habituez pas Cohen une fois le vote lancé normalement, je n'ai pas le droit, mais enfin allez-y. Eh oui, vous n'avez pas le droit, vous me regarder sans rien faire, et puis après vous dites tiens en fait hé ben quoi, je sais qu'il est tard, mais il faut rester réveillé allez Madame Cohen. Ben merci infiniment Monsieur le le le président, simplement je, je pense que c'est important effectivement de de redire, 2, 3 petites choses qui conforte d'ailleurs les propos que j'ai tenus lors de la discussion générale, je je regrette vraiment que, à l'occasion de cette PPL, nous ne nous soyons pas donner les outils pour contrebalancer le le pouvoir des industriels du médicament, on a vu et il y a eu des exemples qui ont été données à la fois au niveau de mon groupe mais aussi sur d'autres bancs du fait que, il y avait des prix absolument exorbitant qui était fixé sur un certain nombre de médicaments dans la plus grande opacité que ça coûte énormément d'argent à l'assurance maladie et que il n'y a absolument aucun contre-pouvoir, donc je pense que l'urgence et surtout à la lumière de ce qu'on vient de vivre au niveau de la la crise sanitaire, c'est d'avoir effectivement un outil qui nous permettent de réguler tout ça et cet outil, c'est effectivement un pôle public, notamment du médicament et c'est aussi le fait de ne pas aller dans le sens des industries du médicament comme le lait, qui ont un gros pouvoir de lobbying et qui influence un certain nombre de, de, de nos collègues et je le regrette tout à fait et c'est pourquoi je le redis ici : si le gouvernement n'a pas de contre-pouvoir, hé bien, la loi est faite par ceux qui pensent à effectivement plutôt faire plus de profits, y compris en période de pandémie sans s'occuper réellement de l'intérêt du plus grand nombre et c'est dommageable. Merci beaucoup, vraiment, Monsieur le Président, juste quelques mots rappelez ou expliquer ce que sera le vote du groupe socialiste, écologiste et républicain, puisque certains points qui ont été en discussion ne sont pas acceptables pour notre groupe de la mort, je l'ai dit en discussion générale le rattachement des au CHU, qui met en danger l'indépendance de ces derniers, nous partageons le constat du manque de moyens de mais l'idée selon laquelle le rattachement de CCP des CHU permettrait un accroissement des ressources semble illusoire, hé bien, au contraire, c'est même Hlinka qui nous la note même dit à l'audition, au lieu de partager les ressources du CHU pourrait tout aussi bien se les approprier au détriment des CPP cette pareille mesure ne paraît donc à la fois inefficace et dangereuse, un autre point sur lequel nous aurions bien aimé pouvoir trouver un accord, c'est celui du prix des médicaments qui viennent d'être évoqués par ma collègue Laurence Cohen, la transparence du prix des médicaments est fondamental pour notre groupe, il est indispensable de prendre en compte dans la fixation des prix, le coût réel de production et les investissements publics en recherche de logement dont il a bénéficié, il était, il aurait été intéressant puisqu'on parle d'expérimentation que l'expérimentation dans ce texte, permettent de élargir à ces critères, l'expérimentation en fait nous estimons inutile et même dangereux de soumettre les recherches en sciences humaines, pourtant sur le domaine de la santé à l'évaluation des comités d'éthique et de recherche, la protection des personnes, l'évaluation du fait de l'étendue des recherches potentiellement concernés comporte un risque d'atteinte au principe de liberté de la recherche aussi au vu de ces éléments, le groupe socialiste, écologiste et républicain ne votera pas ce texte et s'abstiendra. Merci donc cette fois jamais aux voit l'ensemble de la proposition de loi relative à l'innovation en santé qui est. Pour. Qui est contre. Qui s'abstient. La proposition de loi est adopté. Petits. Madame la présidente. Rapidement, Monsieur le Président, soyez rassurée, simplement pour remercier, en effet, ceux qui ont voté ce texte, c'est l'aboutissement d'un travail de depuis plusieurs années sur l'accès à l'innovation, bien évidemment, le texte n'est pas complet et on l'a centrée sur quelques points, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'on peut ne pas être favorable au pôle public du médicament, sans être forcément à la solde des laboratoires et nous avons toujours travaillé lors depuis que nous travaillons depuis depuis 2 3 ans avec Véronique Guillotin avec Yves Daudigny auparavant lorsqu'on travaille sur l'accès aux médicaments, on avait 2 objectifs, hein, celui du patient qui doit accepter le plus tôt possible aux médicaments aussi nous étions toujours attentif à ce que nous disait les chercheurs et les professionnels qui soignent les patients atteints de maladies graves, de maladies rares avec ces médicaments innovants, c'était notre objectif et notre boussole, c'était eux et non pas un lobbying quelconque. Merci beaucoup, madame la présidente, madame la Ministre, mes chers collègues, je vais lever la séance prochaine séance mercredi 23 février à 15 heures pour les questions d'actualité au gouvernement la séance.